La séance est reprise. Bien Madame la Ministre chers collègues nous allons. Reprendre la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuel. Je vous rappelle que la discussion générale est Close. Nous passons donc à la discussion du texte de la commission. Et avant l'article 1er, nous avons un premier amendement. Défendu par monsieur Assouline ou Madame Robert. L'amendement 26. À

C'est un article additionnel avant l'article 1er. Cet amendement tend à consolider une chaîne et une radio du service public comme référence en matière de sport. Cela reprend. Une proposition que j'avais pu évoquer. Dans un rapport. Cet amendement ne reprend une proposition déjà débattu dans le cadre de la loi 2021 relatives à la protection des Oeuvres culturelles à l'ère numérique. Issue de mon rapport relatives à la place du sport à la télévision en France, remis au gouvernement en septembre 2016. À cette occasion j'avais émis le souhait de conforter le rôle de service public dans la mise en valeur du sport à la télévision. Et dégager plusieurs pistes pour atteindre cet objectif, et plus particulièrement celle d'instituer au sein du groupe France Télévision, une chaîne référence en la matière. Les chiffres présentés dans ce rapport sont éloquents. En 2015, France Télévisions avait diffusé un peu plus de 1000 heures de sport. Il s'agit de la seule société capable d'offrir au public une telle quantité d'émissions et de retransmission. Seule la chaîne l'équipe qui est uniquement consacrée au sport assume par ailleurs ce type de retransmission. En août sa couverture multi-chaînes de grands événements sportifs. Tour de France, Rolland Garros Jeux olympiques constitue un atout supplémentaire. Compte tenu des contraintes et des spécificités des différentes chaînes du groupe. J'avais évoqué qu'à l'époque plusieurs pistes à mes yeux un positionnement spécifique ne remet pas en cause la stratégie globale et transversale de diffusion de contenus sportifs mis en place par France Télévisions et n'aurait pas pour effet de désinvestir, France 2 et France 3 de la couverture de grands événements en août cela serait complémentaire avec le développement de France TV, Sport. J'espère donc que le, ça le Sénat aura à coeur d'assurer une meilleure Exposition du sport dans les médias publics en clair et gratuit il conforterait ainsi le rôle Merci. Avis de la commission sur cet amendement. Toutefois il n'apparaît pas judicieux de préciser dans la loi la programmation de chacun des services du groupe public, ce qui reviendrait en réalité à établir un conventionnement par chaîne comme cela existe déjà pour les chaînes privées. Il apparaît au contraire préférable de laisser la plus grande souplesse possible aux dirigeants des chaînes afin de définir l'identité de chaque chaîne, et de pouvoir le, la faire évoluer en fonction des attentes du public, c'est un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur, madame la ministre. Avis du gouvernement.

une complémentarité des chaînes comme on a pu le voir pour le Tour de France pour Roland Garros donc même avis que le rapporteur avis défavorable. Merci monsieur Assouline. Oui bon qu'il n'y a pas de confusion c'est je l'ai dit d'ailleurs c'est pas une chaîne spécifique. Ça ne remet pas en cause le fait que c'est. Ça doit être transversale. Mais une référence. Une chaîne référente. Tout, on était bien dans des équipes, ce que veut dire référente. C'est-à-dire qu'il y a un rôle un peu de pilotage de de de de. De de de distribution des rôles, et qui permet de. De fidéliser. Le téléspectateur sur une chaîne pour un certain nombre d'événements qui ne trouvera pas ailleurs. De toute façon. Le sujet que j'évoque là. C'est un sujet qui va revenir dans notre dans nos débats parce que on ne pourra pas esquiver le fait que. Le service public. Qui remplit cette mission déjà de diffuser des sports que personne ne diffuse. Est évincé. De tous les sports. À grande audience. Parce que les droits. Sont beaucoup trop cher pour le service public et qu'en général ces manifestations qui ont lieu après 20h. Eh bien quand on n'a pas la publicité pour se payer. Ces manifestations. On est à tout de suite, au point que. France Télévisions a du mal à se positionner sur quelque chose qui serait complètement dans sa vocation, l'équipe de France féminine. Qui va participer au Mondial. J'entends que avec M6. Il a une offre qui va être fait, mais en tous les cas on ne peut pas accepter cette situation trop longtemps j'ai d'autres propositions. Nous avons d'autres propositions à faire pour pour que France Télévisions et le service public se positionne sur les manifestations sportives un grand public parce que même celle qu'elle a aujourd'hui comme Roland Garros, vous avez vu qu'Amazon a déjà grignoté et que il faut faire cesser cette dérive. Merci donc je vais soumettre aux voix. Cet amendement. Qui est avec deux un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Au drame Mandement avant article additionnel avant l'article 1er Madame de Marco. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Après la suppression de la contribution à l'audiovisuel public dans la loi de finances rectificative 2022 le Conseil constitutionnel mis une. Un avis de réserve de constitutionnalité destiné à garantir l'affectation des ressources suffisantes pour les sociétés publiques en fait qu'elles puissent contribuer de poursuivent leur mission de service public. Dans le souci de garantir des ressources pérennes pour l'audiovisuel public. Cet amendement reprend une proposition faite. Lors de la commission d'enquête sur l'indépendance des médias. Il vise à instaurer un crédit d'impôt pour l'acquisition de bons émis par une société audiovisuelle public. Il s'agit également d'une proposition de l'économiste Julia KG qui a inspiré la proposition de loi Fortesa et orphelins en 2022 à l'Assemblée. Cela correspond à la volonté de rendre le citoyen auditeur plus actif dans son soutien aux médias enfin de renforcer son indépendance. Le montant maximum, établi à 150 euros se situe entre le montant de l'ancienne redevance à 30 138 euros et le prix de l'abonnement de NEC suisse à 14 euros par mois environ. Pour le contribuable. Il s'agit d'un mécanisme fiscal plus acceptable que ce n'était la contribution à l'audiovisuel public. Faute de progressivité, il renforce le consentement à l'impôt à une période où l'inflation baisse. Le pouvoir d'achat. Il peut s'agir ne voit de réaffectation comme la piste une contribution progressive. Voilà cette piste devrait être explorées. Merci cher collègue. À monsieur le rapporteur. Pour la commission. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à créer un crédit d'impôt pour inciter les Français à financer l'audiovisuel public. Il ne fixe cependant aucun objectif en termes de crédits attendu. Pardon. Et ne propose aucune évaluation du coût du dispositif pour les finances publiques. Il apparaît plus urgent de clarifier le financement de l'audiovisuel public de son organisation et de sa gouvernance avant d'imaginer un autre dispositif qui ne pourra jouer qu'un rôle marginal dans le financement de l'audiovisuel public. C'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Monsieur le président, avis défavorable également même si je comprends l'esprit de votre proposition pour qui est aussi une adhésion encore plus forte des citoyens, mais quant à l'indépendance. Je suis le public, elle est déjà garanti nomination des dirigeants par l'Arcom et non par le gouvernement totale indépendance éditoriale. Et je ne suis pas sûr que cette proposition vise réellement à à. Garantir encore plus l'indépendance avis défavorable. Bien merci donc un double avis défavorable je vais soumettre l'amendement on voit qui est enfin Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons la discussion des amendements sur l'article 1er. Donc nous avons quatre amendements discutés identique en discussion commune. Le premier monsieur Bargeton. Merci Monsieur le Président bon rentre dans le sujet dans le vif du sujet de de la Holding. Je serais peut-être plus court après c'est aux autres amendements parce qu'ils sont tous évidemment cohérent et sans avec les autres partir du moment où je propose un amendement de suppression. L'article 1 an je je propose ensuite les amendements de suppression de de la suite alors. Le seul Avantage d'une d'une Holding, c'est que ça, ça ferait travailler les cabinets privés, moi je, j'avais cru comprendre qu'il fallait arrêter de le faire c'est sûr que il va falloir mouliner hein pour le mettre en place

la vue de la fusion. L'idée de cette Holding par rapport à ce que vous pensez, on a l'impression que vous vous arrêtez un peu au milieu du gué et que il y a une forme d'ambiguïté. Par rapport à une solution qui d'ailleurs d'après vous selon vos, vos, vos propres. Vos préoccupation pardon. Finalement présenterait les avantages sans avoir les inconvénients parce que le risque d'une Holding, on le sait, c'est que ça coûte de l'argent, puisque vous rajouté une strate et qu'on supprime pas le reste en réalité ça ça peut arriver en France, on a des exemples de, de rapport là dessus je reviens pas sur certaines critiques qui ont pu être formulées à pour telle ou telle réforme c'est c'est rajoute une strate et on supprime pas et donc en fait ça rajoute du cou et de la bureaucratie supplémentaire, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps au détriment de l'action. Des dirigeants. Au service de de de leur objectif. Ça pourrait retarder les les contrats d'objectifs et de moyens qui doivent être renouvelés en 2024 2028, donc ça va plutôt freiné retarder des mutualisations qui sont en cours et voie d'approfondissement et puis. Ça ne répond pas à tous les enjeux qualitatifs qui sont plutôt le rajeunissement de l'audience, l'accélération de la transition numérique. Donc au fond, vous auriez pu avoir le courage d'assumer jusqu'au bout. Votre radicalité. Bien merci. L'amendement numéro 12 monsieur Assouline. Puis on reviendra pas plusieurs explications mais. Très franchement. C'est une proposition, on dirait que c'est comme une marotte parce que. Bien entendu que c'est quelque chose qu'on pouvait discuter autrement en 2015. À l'époque il y avait très peu de synergies. Mais notre débat servi. Et des positions du Sénat ont servi parce que depuis ça impulsé ça a poussé à l'intérieur même des sociétés Radio France où il y a plusieurs radios de Radio-France à travailler ensemble. À France Télévision les chaînes différentes. Des efforts énormes des salariés parce qu'on ne les oublie souvent et en terme d'investissement parce que c'est à chaque fois. Hé bien un esprit pionnier, qu'il faut pour reconstruire une façon de travailler. Et ils l'ont fait et il faut les féliciter. Un prix à payer. 4000. Et quelques en. Équivalent temps plein. D'emplois supprimés donc. À Radio France avec sa plus longue grève de son histoire. France Télévisions, qui avait déjà essuyé plusieurs plans de plusieurs milliers de personnes, c'était encore 900 emplois supprimés Dans un tel paysages dire que bah. Malgré ses efforts, malgré ces synergies malgré les résultats il y a des résultats, tant dans le numérique dans l'invention regarder Radio France. Il détrône toutes les autres radios alors qu'on les avait enterrés. Malgré une qualité de programme, notamment dans l'investigation à France Télévisions une quelque chose de plus. Malgré tout cela on dit en fait que tant qu'il y a un salarié à France Télévisions. Il est trop. C'est ça qu'on leur dit qu'on leur envoie comme message au lieu de les applaudir et de les encourager et puis. La Holding aujourd'hui ne permet pas de rationaliser. Car nous savons que ce sera entre 20, 30 à 50 millions le coût supplémentaire pour l'audiovisuel public et donc l'inverse de ce qui a l'air d'être. Voulue par les auteurs de la loi. Le drap sur d'autres arguments ensuite. Merci monsieur Assouline Monsieur Bakhit. Merci monsieur le président, madame. Les ministres, mes chers collègues, quelques mois après la suppression de la redevance et une fois de plus le service public de l'audiovisuel et questionné dans son offre mais aussi dans son modèle, un bilan des dynamiques des médias publics plutôt positif comme je le soulignais tout à l'heure dans mon intervention le changement coopérer cette Holding risque de créer une nouvelle inertie des institutions un public visé pourtant doivent. Auquel doivent nos entreprises publiques audiovisuelles sont immenses numérisation reconquérir le public adolescents et jeunes adultes. Lutter contre la désinformation et les infox mobiliser les forces vives de notre service public un projet bureaucratique qui ne colle pas avec la diversité que représentent les métiers et savoir-faire incluse dans l'audiovisuel public d'abord. Parce que les modalités de désignation de cette Holding ne présente pas les garanties suffisantes au maintien de son indépendance et ensuite le pouvoir accordé au directeur général de la Holding en matière de choix dans la répartition des Budgets entre les différentes entités fait craindre au regard de l'objectif mise en avant de la Holding de concurrencer notamment les plateformes. Que la radio, je le disais aussi, soit le parent pauvre de ce futur audiovisuel. Par conséquent, le risque de cette Holding, c'est de supprimer toute obligation en matière diversité cette Holding qui a l'intention de défendre le service public de l'audiovisuel va en réalité dans la pratique détériorée, selon nous un peu plus les Budgets des filiales déjà largement érodé, je vous remercie. Merci monsieur le président. Donc la proposition de créer cette Holding rassemblant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l'Institut national de l'audiovisuel n'est pas souhaitable. Cette proposition ne repose notre sang sur aucune justification valable y compris budgétaires. Nous avons le recul pour savoir qu'une telle hypothèse aurait pour conséquence d'accroître les coûts de fonctionnement. Et l'inquiétude également des salariés. Derrière ce projet de Holding. Il y a bien sûr la volonté d'ouvrir la voie à de nouveaux plans de restructuration. Cela n'est pas sans risque pour le pluralisme, la diversité Lekto électorale, l'identité de RFI par exemple complètement dissous tous autour de au sein de France Médias Monde et les salariés de Radio France craignent la marginalisation de leur média ou au musée, fils de contenus visuels. Or il s'agit du média le plus accessible pour toutes les catégories de la population. Le journalisme et la production audiovisuelle de qualité ont un prix, il est nécessaire de renforcer donc le journaliste de terrain. Les équipes d'envoyés spéciaux pas les technos scrutin. C'est pourquoi nous nous opposons à cette Holding. Bien merci chers collègue monsieur le rapporteur. Avis sur ces quatre amendements de suppression. si vous me le permettez j'j'aimerais revenir sur le un argument souvent mis en avant sur le coût de la Holding. Le débat sur le coût de la Holding est un faux débat puisque, selon la présidence de France Télévisions elles-mêmes aucune étude n'a été faite sur le sujet. L'argument vise donc avant tout à défendre le statu quo, quand bien même celui-ci risque d'être fatal pour l'audiovisuel public. Le président font a toujours défendu l'idée d'une structure souple Les auditions que nous avons menées ont montré que ça l'a été possible compte tenu des grilles de rémunération que nous avons. Obtenues. Sur une équipe de d'une vingtaine de personnes, cela peut correspondre environ à 3 millions d'euros. À noter que la majeure partie de ces personnes travaillent déjà dans les entreprises considérées. Il s'agit donc d'un coût brut et non d'un coup net. Ces 3 millions doivent représenter mais je prends cet exemple là à à peu de choses près excusez cette. Légère imprécision. Mais c'est exactement le montant des hospitalités que vient de dépenser France Télévisions lors du festival de Cannes et je n'ai entendu personne dans cet hémicycle dénoncer cette dépense qui n'était peut-être pas tout à fait indispensable. J'ajoute que la nomination d'un responsable unique de la stratégie ayant la possibilité de trancher enfin les différends entre les filiales fera économiser beaucoup de temps et d'argent avec cette gouvernance France Télévision n'aurait pas eu besoin de savants tué par exemple dans Salto en perdant 80 millions d'euros, car un agrégateur de contenu, de l'ensemble de l'audiovisuel public existerait depuis des années la chaîne FranceInfo aurait été développée de manière attractive sur la base de France 24, l'offre de proximité serait déjà une réalité. En somme, l'audiovisuel public du futur ça déjà depuis longtemps une réalité. Madame la Ministre. Merci monsieur le président. J'ai eu l'occasion de de le dire lors de la discussion générale. Je ne vais pas redéployer. Tout ce que j'ai, j'ai indiqué, je suis favorable aux amendements de suppression puisque je suis défavorable à la création de cette Holding oui à une nouvelle ambition pour les 5 prochaines années pour le diésel public oui pour le traduire dans les contrats d'objectifs et de moyens en renforçant les coopérations et le suivi de ces coopérations. Oui pour plus de souplesse, de concertation. D'avancées pragmatiques et ambitieuses mais non à la bureaucratie non lourdeurs d'organisation et non à une strate hiérarchique qui viendraient ralentir. Les et dispersé les énergies. Merci. Monsieur le Président la font. la le débat c'est, est-ce qu'on continue à partir des comme où on est insatisfait des comme et on essaye de passer à une autre organisation qui permettra d'aller plus loin, plus vite sur les coopérations entre les deux, entre les La Holding pourquoi nous la proposons parce que maintenant nous avons du recul sur l'efficacité ou devrais-je dire l'inefficacité des comme et, c'est pas nous qui le disons, c'est pas un point de vue subjectif c'est l'Arcom qui est chargé de justement de, de contrôler, c'est comme qui le dit très bien dans son avis du du 15 janvier 2021, le CSA avait regretté le manque d'ambition de ces derniers en matière de synergie au sein de l'audiovisuel public et l'absence de structures du pilotage coordination de de chantiers comme je cite encore, la coopération au sein de l'audiovisuel public demeure limitée et la convergence TV, radio et très en deçà de la situation d'autres services publics européens et les faits malheureusement le sont.

ouf ou font l'objet ont fait l'objet d'une mutualisation sur les formations mutualiser, elle ne représente que 2% à France Télévisions et 5% pour Radio France, sur les matinales communes France 3, France Bleu. Prévu initialement pour une généralisation en 2022 l'objectif n'est pas atteint et elle n'est pas, il ne sera pas atteint au mieux avant 2025. D'après Philippe partie des directeur du réseau régional de France 3 et enfin sur les marchés qui ne vous devrait nous permettent de faire des économies, c'est des choses réelles et qui supporteront largement le coup de de la Holding. Holding. Je je cite il est marginal, comme le note l'Arcom dans son rapport de fin 2022, seulement 40 marcher groupées pour un montant cumulé, tenez-vous bien, de 45 millions sur un chiffre d'affaires, une activité globale de plus de 3 milliards et demi, on voit bien que les comme ne fonctionne pas. Alors bien sûr on peut se satisfaire des annonces au moment de la. La négociation et de la signature de ces comme mais il faut maintenant avoir la lucidité de regarder le résultat et le résultat n'est pas bon. Président Karoutchi. Oui, monsieur le Président Madame la Ministre moi je d'abord je suis admiratif. Sur le plan politique c'est j'allais dire. Taux a fait des émules. Parce que franchement quand j'entends notre collègue Bargeton Madame la Ministre dire comment comment. Mais quelle horreur. Une solution bureaucratique. La création d'une Holding. Mais qu'est-ce que vous imaginez à droite. La Holding, c'était dans le projet de loi du gouvernement. Riester, votre collègue au gouvernement, il y a 3 ans, donc j'en déduis que c'est peut-être pas chez nous que d'un coup quelqu'un s'est dit pourquoi pas une Holding la la Holding, c'était l'idée qui circulait dans les milieux gouvernementaux dans les ministères et dans une partie de cet hémicycle il y a déjà 4 ans. Donc en la matière. Il faut rester quand même un petit peu cohérent par rapport à ce qu'on a débattu, est ce qu'on a déjà dit ici et pour reprendre ce que vient de dire le président la font. Si les convergences parce que ça on nous l'a beaucoup dit, mais si les convergences avait magnifiquement fonctionné depuis le temps qu'on en parle depuis 7 8 ans. Si les convergences étaient. Évidente moi personne ici ne viendrait dire, ni fusion ni Holding ni quoique ce soit, on se dirait ben c'est très bien, les résultats sont probants dans les convergences avançons continuons d'avancer à ce rythme et on va avancer tranquillement le le problème c'est que tout le monde, pas seulement l'Arcom. Mais même quand on auditionne les responsables de l'audiovisuel. Ils vous disent même c'est vrai que en domaine dans le domaine de la convergence. On devrait faire plus, on devrait faire mieux ben voilà le problème c'est qu'au bout de 7 8 ans il y a pas les résultats attendus en matière de convergence donc soit on ne change rien et c'est un signal pour tout le monde y compris pour les acteurs de dire ne vous inquiétez pas. Aucune modification de structure donc continuer sur le rythme actuel et je crois que la notion même de Holding doit permettre de peut être secoué un peu le cocotier pour que les choses bougent. le problème c'est que la Holding. Ce n'est pas une notion pour secouer le cocotier. C'est une réalité. Donc, projetons-nous sur sa réalisation. Bien entendu que tout ce que vous pointez, on peut faire mieux, c'est insuffisant et tout OK. Le problème c'est que l'outil Holding ne répond pas aux difficultés rencontrées. Donc si on se projette c'est quoi. Hé bien, demain il y a une réorganisation complète de toutes ces sociétés. Et toute l'énergie, la tension, les conflits sociaux. Vont être portés sur comment se réorganise, avec les guerres internes, avec les guerres de pouvoir avec les instabilité pour les personnels, avec les craintes des fois pas justifier des fois justifié. Alors que on doit maintenant justement pointé là où il y a des avancées à faire et poussé et que l'ensemble des personnels soient tournés vers une seule chose, la qualité de ce service public la qualité des émissions et des programmes proposés. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu, c'est une attention permanente dans le monde des médias. Si on s'effondre, un jour on reprend papier. Vous savez, il se médiamétrie tous les jours il y a les audiences qui tombe et. Donc il y a une mobilisation extraordinaire de tous les personnels dans ces chaînes et dans ces radios pour être à la hauteur tenir parce qu'il y a les Gafam, d'un côté parce qu'il y a la concurrence privée totalement légitime et que il faut tenir son rang. Donc vous voulez aujourd'hui qu'on dise toute cette énergie va t'as une réorganisation est ce que ça vaut le coup si tout s'effondrer, si la qualité des programmes étaient pas bonnes, si il y avait moins de 10 maths on dirait OK de toute façon il faut une thérapie de choc mais aujourd'hui. La thérapie de choc pas ce sera ça la Holding. Dans sa concrétisation aujourd'hui viendra au contraire désorganisé et et démoraliser les personnels et faire en sorte que l'attention au public soit la dernière roue du carrosse. Or, ça doit être le premier. Rapidement monsieur le président. Depuis 2020, comme le contexte a changé. Une forme de pression, une forme de. Le débat a prospéré et le fait que deux dirigeantes par les moindres Delphine Ernotte et Sybille veulent se soit prononcée en février 2023 pour un plan stratégique unique avec des propositions d'objectifs communs de socle de travail à proximité et cetera, ça n'est pas rien non plus le fait que il y ait un socle commun à l'ancien à l'ensemble des contrats d'objectifs et de moyens. Pour aussi faire confiance à un moment aux acteurs quitte à à trouver des des des moyens pour que pour vérifier pour évaluer davantage et s'assurer que les coopérations soit vraiment renforcer mais on peut faire confiance aux acteurs qui ont changé de discours et de postures par rapport à des, à des coopérations parce qu'elles ont aussi ces sociétés compris qu'elle devait. Aller plus vite. Accélérer et renforcer cette coopération et ces. Mutualisation, donc c'est quand même un point important, je crois qu'il faut souligner un peu de de pragmatisme en l'occurrence ne nuit pas par rapport à une soupe à une solution qui ne répond pas à des problèmes qui sont très concrets. Rajeunissement des audiences, c'est pas une question de Holding c'est de rajeunir les audiences. Merci cher collègue donc. Il n'y a plus de prise de parole Madame Morin-Desailly pardon. quelques mots pour. Apporter un peu d'éclairage au débat qui est très importante puisque la création de cette Holding. C'est au coeur de la. Proposition de loi, ce n'est pas parti de rien, cette idée de J'ai voulu le dire dans le propos liminaire. À la tribune, ça résulte d'un travail de fond extrêmement. Important qui a été réalisé depuis des années par notre commission avec une convergence de vue. Idée qui était déjà un peu dans les tuyaux en 2009 quand on a pris conscience qu'avec la transition numérique on aborderait en fait la question des publics non pas en silos en vantant toujours chaîne par chaîne groupe par groupe Programmation audiovisuelle mais désormais pas porte d'entrée thématiques. David Assouline à juste titre réclament une meilleure lisibilité pour le sport moi je partage complètement cette ambition mais je sais. Pas sûr aujourd'hui que c'est une chaîne du sport dédié qui est la bonne porte d'entrée. Je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt l'objectif de se dire le. Sport et transversale. On a des commentaires sur le sport à la radio, on a la les les manifestations. Sportives de proximité qui sont reliés par les chaînes de France 3 et de France Bleu. On le voit bien tout le week-end dans nos propres. Départements. On a les grandes manifestations sportives nationales, internationales, c'est sûr. L'idée c'est, c'est de rendre lisible et cohérent et enrichit mutuellement cette porte d'entrée généraliste sur le sport et c'est pas en stylo c'est de manière transversale et je pense que la Holding c'est comment dirais-je infuser cet état d'esprit que désormais on doit travailler par thématiques, France Culture, France Médias sera France Culture, France Info. Eurosport France, jeunesse, la thématique du régiment de la jeunesse, ça doit être l'objectif partagé et on est tous en ordre de marche donc. Pour rajeunir et faire les investissements qui vont ensemble de manière stratégique, et je pense que pour aller plus loin dans les coopérations, il faut quand même un chef d'orchestre. Je le pense très sincèrement, non pas pour décourager les personnels, c'est au contraire pour les mettre tous sont en de marge pour. Pérenniser leur modèle, c'est pas pour rien si l'ensemble des audiovisuels publics européens ont fait leur mue depuis longtemps vers ce modèle donc réfléchissons à cela quand même regarde autour de nous. Richard Koller merci. Madame la ministre. Merci monsieur le président, en, en quelques mots. Pour aussi indiquer que tout ne passe pas par des convergences. On le sait certaines. Priorités vont nécessiter des coopérations accrue. Les entreprises y sont prêtes, font des propositions très concrètes. Je pense notamment à la lutte contre la désinformation qui a un enjeu absolument crucial et le premier pour moi. Mais dans d'autres domaines, par exemple sur le numérique, le digital. On sait très bien et on l'a vu. De ce qui se passe chez nos voisins européens. Les plateformes Audio et vidéo sont séparés. Même la BBC a re séparer les plateformes Audio et vidéo Toutes les priorités ne passe pas par des coopérations, des convergences ou des fusions. Donc il faut bien aussi scinder les sujets. Qu'on ait une ambition sur quelques chose. Autoritaire, il me semble que toutes nos discussions ces derniers mois montre au moins que nous sommes d'accord largement sur ses grands enjeux sur les créations sur la jeunesse sur le numérique sur l'information et sur la proximité. On a bien vu que FranceInfo a pu se faire sans Holding ici la plateforme France 3, France Bleu. Ce fait sans la Holding et avance certes. Ça peut aller plus vite mais tout de même ça avance les synergies mobilières, on sait très bien que ça prend énormément d'années quel que soit le schéma. Donc les les projets de coopération quand elles sont justifiées, quand elles sont comprises, quand elles sont. Portées par les équipes avant sans qu'il ait besoin de réorganiser et vu l'accélération depuis 3 ans de la désinformation des phénomènes. De de d'hégémonie des plateformes. je pense que maintenant, l'urgence elle est plutôt d'approfondir les coopérations telles qu'elles sont lancées et nous avons les moyens de renforcer dans les contrats d'objectifs et de moyens ce. Ce suivi des, des coopérations plutôt que de mettre toutes ses énergies dans une nouvelle organisation. Et dans un schéma de mécano institutionnel qui va nécessairement prendre énormément de temps, on sait très bien qu'en France Télévision est devenue France Télévision le nombre d'années qu'il a fallu pour créer une Holding puis une fusion, c'est entre 9 et 12 ans. Est ce qu'on veut prendre ce temps pour ce mécano institutionnel ou est-ce qu'on veut prendre ce temps pour avancer sur les priorités sur lesquelles nous sommes d'accord. Voilà, merci.

Qui est contre. Qui s'abstient. Ou qu'ils ne sont pas adoptés. Je passe à l'adoption de l'article 1er qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté sur l'article 1er bis, un amendement de Madame DeMarco. Pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment. Cette interrogation n'est pas souhaitable afin de laisser à cette chaîne tous les moyens de remplir ses missions spécifiques dans toute la francophonie. TV5 a été créé en 1984 afin de matérialiser l'unité linguistique rassemblant les flaques francophones à travers le monde et constitue un opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Son capital se partage entre les sociétés audiovisuelles publiques françaises belges que suisse canadienne et monégasque au lieu la délimite déjà évoqué de la Holding se pose la question juridique du respect des droits des autres actionnaires de TV5 Monde, a pris une intégration unilatérale de la part française au du capital de la Holding et visait à rappeler aux autres gouvernements bailleurs de TV5 Monde. L'engagement de la France dans le financement de la chaîne francophone internationale, elle est très attendue par la direction de la chaîne qui est venu nous le dire en audition. C'est la raison pour laquelle je demande un avis défavorable. Madame la ministre. Merci monsieur le président. Même avis que le rapporteur avis défavorable. Donc un double avis défavorable je soumets l'amendement voix. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté, je mets aux voix l'article 1er bis qui est pour. Qui est contre.

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement trois que j'avais déposé c'est la composition en capital. La détention par l'état de la Holding. Donc comme j'ai proposé la suppression de la Holding. Je propose la suppression également de cet article Monsieur Assouline ou Madame, Robert celui qui vise à prévoir la nomination des commissaires du gouvernement dans chacune des sociétés de la Holding cette police civilité existe également pour les sociétés dans lesquelles l'État dispose d'un représentant et dont il détient au moins la moitié du capital ces commissaires n'ont qu'une voix consultative sauf dispositions légales contraire ici heureusement non prévues bien sûr dans les conseils d'administration auxquels ils assistent. Néanmoins, il s'agit ici encore de renforcer la mise sous tutelle de l'audiovisuel public par la présence de commissaire du gouvernement dans les CA de chacune des sociétés pas moins de 5 administrateurs nommés par l'État au sein de la Holding sans compétence précise requise. Bon il y a le président en plus donc la moitié des membres et de dans les CA des 4 sociétés sous tutelle. À quoi serviront ces commissaire du gouvernement, si ce n'est ah renforcé de mon point de vue la pression de l'État au des team au détriment de l'objectif de l'indépendance des médias et des rédactions. Donc c'est un amendement important qui bien sûr vient en cohérence avec celui qu'a présenté mon collègue merci. Merci Monsieur Bakhit. Merci monsieur le président, donc créer une super structure réunissant des entités dans la production des programmes et les métiers répondent à des réalités et à des missions très différentes alourdirait considérablement le fonctionnement du service public de l'audiovisuel, comme je l'ai dit, une telle mesure serait aussi budgétivore. Cette mesure est inutile puisque les entreprises de l'audiovisuel public coopère déjà ensemble mais ces coopérations s'amplifie. Je veux, j'en veux pour preuve la création de France TV ou encore d'ici qui sont tous deux le résultat de coopération fructueuse entre France TV Radio France pour ce qui est des mutualisations informatique envisageable. Celles-ci peuvent être tout à fait envisager sans la mise en place d'une Holding par exemple l'initiative de club Data animé par Lina doit bientôt voir le jour en réalité votre proposition ne va qu'alourdir la structure de l'audiovisuel en mettant en place un étage des ici Lionel supplémentaire qui ne présage rien de plus que des années d'Ibos, milices malheur ou l'évolution rapide de ce secteur nécessite au contraire l'agilité de l'adaptabilité, mais aussi et surtout de la rapidité décisionnelle. Je vous remercie. Merci et Madame de Marco. Merci monsieur le président comme les autres dispositions du titre 1er. Nous nous opposons à cette disposition en apparence protectrice pour l'audiovisuel public français. Il s'agit en réalité de l'heure puisque la détention intégrale du capital de la Holding par l'État ne constitue en aucun cas une garantie de maintien d'un niveau satisfaisant de ressources, a fortiori lorsque le même texte prévoit la possibilité de revoir les conventions stratégique pleurer. Pluriannuel avant leur terme. Merci. Avis de la commission sur ces quatre amendements. C'était déjà dans le projet de loi Riester par, j'allais dire presque coordination avec la loi de 86, donc je le le l'argument sur le fait que ça serait nouveau et ne ne tient pas. Voilà, avis défavorable. Madame la Ministre. Monsieur le président. Avis favorable aux amendements de suppression en cohérence avec ce que j'ai dit précédemment. Bien merci monsieur Assouline. Non mais c'est. Cohérent. Peut être avec la loi Riester mais c'est pas cohérent avec les principes qui juste. Dicté un petit peu la façon dont tu n'appréhender. La gouvernance du service public et les débats qui ont pu avoir lieu, parce que là de quoi il s'agit. On a un PDG. On va voir comment il est nommé je vois que le rapporteur a changé son fusil d'épaule sur le mode de nomination et qu'il a entendu ce que nous le proposions par amendement en anticipant et en faisant sauter une autre mais on en parlera tout à l'heure. Mais. Ensuite, il nomme des directeurs. Ensuite il y a plus de comme par société. C'est lui qui décide. Les sommes versées à chaque société jusqu'à présent, y compris nous parlementaires. On avait un avis à donner sur chaque homme et aussi sur chaque ligne budgétaire. C'est fini. Donc c'est la fin et d'un contrôle parlementaire. Mais ça fait triompher quelque chose que je pensais pas que ça viendrait des républicains. Une gestion très bureaucratique qui viendraient. D'en haut et qui viendrait douter de l'initiative et de la souplesse. Et je suis heureux d'ailleurs que ce soit communiste, qui a plaidé pour l'agilité, la souplesse, face à la bureaucratie que nous proposent les républicains. Oui les, les temps changent et en tous les cas. C'est bien. Que les débats puisse évoluer dans ce sens. Je ne comprends pas. Que vous ne voyez pas où est le problème avec ce mode de gestion. L'usine à gaz que vous créez. La perte de contrôle du Parlement et. Le bridage de l'indépendance de l'audiovisuel public vis-à-vis du pouvoir politique, ça vient en contradiction, d'ailleurs Monsieur Bonnet avec tout ce que vous avez dit dans la commission d'enquête en disant que le service public était à la botte du pouvoir qu'il fallait arrêter avec ça, hé bien. Vous en prenez pas le chemin dans vos propositions. Bien merci monsieur Assouline. Donc nous allons passer au vote sur ces quatre amendements avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 2. Qui pour l'article 2. Qui est contre. Il s'abstient-il être adopté. Nous passons à l'article 3. Et nous avons là aussi quatre amendements de suppression monsieur Bargeton. Défendu. Monsieur Assouline ou Madame Robert. Moi je suis souligné. Alors par cet amendement. On demande la suppression de l'un des articles phares concernant la Holding celui disposant de sa gouvernance et du mode de désignation des membres des conseils d'administration. Je viens d'en parler de façon générale. Exit l'indépendance de chacune des 4 sociétés concernées. France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA Arte. Grâce aux traités qui lient la France à l'Allemagne et TV5 Monde, par le fait que son capital n'est pas détenue intégralement par la France. Exit les présidents de chaque société de simples directeurs généraux. Des 4 sociétés seront placées sous tutelle un président de la Holding tout tout puissant n'assumant que les tâches ingrates ou potentiellement à risque, gestion des mouvements de grève et il risque d'y en avoir, suite à cette réforme d'ailleurs, directeur des publications. Par dérogation au droit commun des médias. Quant au super président directeur général de France Médias. Il sera à nouveau nommé par décret en Conseil des mini-sur proposition. Non Il ne le sera plus que comme initialement prévu. En débat en commission puisque nous avons appris tout à l'heure, en réunissant la commission que le le rapporteur accéder à notre demande. Sur le mode de nomination. Et c'est bien maintenant l'Arcom comme vous le souhaitez. C'était une avancée de la loi sur l'indépendance du service public de l'audiovisuel de 2012. 2012 2013 le c'est plus. Que nous avions initié la gauche à ce moment-là pour arrêter avec un mode de domination qui était celui mis en place sous Nicolas Sarkozy. Je me réjouissais des bruits qui couraient de dépôt d'amendements de la part de la majorité. Sur ce mode de nomination. Je suis content que ce débat soit derrière nous et que. Même si ce n'est pas satisfaisant sur ce mode de nomination. On a été entendu et le danger a été vu. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, nous proposons la suppression de cet article 3 qui effectivement décline la gouvernance de cette Holding et notamment la nomination par le PDG de la Holding des différents directeurs des entités qui la composent. Nous nous y opposons parce que. Il semblerait. Ici que soit mis en avant le fait que la création d'une Holding et est ce que vous appelez des synergies soit la réponse. À peu près tous les. Toutes les difficultés de tous les enjeux qui se présentent à l'audiovisuel public. Or un des enjeux. Qui devrait nous faire réfléchir les uns et les autres, c'est précisément d'assurer la qualité d'assurer la diversité. c'est d'assurer des financements pérennes. Vous avez l'air très tranquilliser Madame la Ministre sur la pérennité des financements de l'audiovisuel. On voit bien à travers cet article que le PDG aura la main sur la répartition des fonds entre les différentes entités. Es dans un contexte où à nos yeux la pérennité financière n'est pas garantie parce qu'elle n'est pas de la même nature. Lorsqu'on a des financements qui sont données par l'État que lorsqu'on avait. La redevance que Jack Ralite se plaisait à appeler une forme d'actionnariat populaire

qui pourrait être le parent pauvre de cette répartition, on pourrait évoquer des tas d'autres sujets et donc il nous semble que cette gouvernance. Y compris quand on la prend un peu plus en détail que la Holding d'une façon générale pose de nombreux problèmes. Merci et Madame de Marco. Merci je vais compléter. Comme les articles précédents. Cet article relatif aurait gouvernance au sein de la Holding ne nous satisfait pas. La complexité des articulations juridique entre les rôles de président de la Holding et c'est des directeurs de chaque société laisse à notre sens présager des difficultés à venir. Celle-ci risque le de prendre le pas sur la coopération et des synergies. Et je dirais il est probable que le rapidement le président nouveau président considère que pour prendre une décision, il faut être nombre impair de personnes et que trois, ce sera déjà trop. monsieur le rapporteur. Sur ces quatre amendements. Merci monsieur le président. Comme ce sont des articles de suppression. Il n'y a pas de d'étonnement à ce que ça soit un avis défavorable. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'expliquer le nouveau dispositif prévu à l'article 100. Madame la ministre. mais. Encore une fois nous avons compensé à l'euro près. Le financement qui était le même que la contribution à l'audiovisuel public, compenser les effets fiscaux. Nous avons déjà eu ce débat la redevance en elle-même n'était en rien une garantie de l'indépendance en tant que telle. L'indépendance, encore une fois, elle vient du mode de nomination des dirigeants qui aujourd'hui. Fait par l'Arcom, l'ancien c'est ça. Elle vient d'indépendance éditoriale, qui est totale et j'y suis absolument attachés. Merci. Bien, donc avis défavorable de la commission. Avis favorable du gouvernement. Je mets les amendements voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés nous poursuivons l'examen des amendements sur l'article 3 avec un amendement de monsieur Assouline le 27. Oui, alors c'est un amendement numéro 27 est inspiré de des 32 propositions de la commission d'enquête. Sur la concentration dans les médias. on avait imaginé. Pour le secteur privé. Que dans tous les conseils d'administration, il fallait. Un administrateur. Qui puisse être là. Pour. Disons, veiller à l'impartialité. À l'indépendance de l'information. Je me souviens que Monsieur Suspicieux du service public. Disait oui vous faites ça dans le privé, mais regardez. Le public, moi je ne dis pas de problème. On peut généraliser et faire que dans l'ensemble, les conseils d'administration. Il y a un tel administrateurs garant de l'indépendance. De l'information garant qui n'est pas d'ingérence. Sur les contenus proposés et donc. Puisqu'on parle de l'audiovisuel public. Je propose avec mon groupe de prendre sa proposition. De la commission d'enquête sur la concentration dans les médias et de vous l'a proposé ce soir. Merci à vie de monsieur le rapporteur. Monsieur le Président l'impartialité de l'information sur les antennes du service public, constitue l'un des fondements de son identité et de sa légitimité. Pourtant elle ne figure pas aujourd'hui parmi les critères qui s'impose aux antennes publiques selon les termes du 4ème alinéa de l'article 43 11 de la loi du 30 septembre 86 et aucune autorité n'est par conséquent chargé de veiller à son respect. Ce qui crée des polémiques qui porte un préjudice évident au service public et affaiblit sa légitimité. L'amendement proposé par notre collègue David Assouline apporte un élément de réponse pour garantir l'impartialité de l'information sur le service public. Il me semble important d'y apporter notre plein soutien. C'est un avis favorable. commenter chaque amendement concernant la composition du CA donc demande de retrait. Monsieur Assouline. Oui c'est. C'est pas l'attitude que vous allez avoir tout le temps puisque vous dites favorables ou pas sur des amendements, alors que vous êtes contre cette loi globalement et et vous êtes contre la Holding mais bon c'est c'est pas grave je je je veux juste. alors pourquoi parce que nous aussi nous sommes pour la suppression de la Holding et on propose des débats. Parce que de toute façon derrière on votera raconte l'article. On propose des débats et un des débats, c'est celui de. Penser, et d'ailleurs je le pense en projection parce que c'est dans les grands groupes privés qu'il faudra aussi se battre pour cela parce que c'est là où on a constaté dans la commission d'enquête des ingérences évidentes. J'ai encore lu un article dans le monde. Le la semaine dernière qui relate la fin du processus de prise de Lagardère par Bolloré et y compris. Ça, ça touche, Bernard Arnault et. et. Qui nous ont dit dans la commission d'enquête que jamais au grand jamais s'ingérer. On a l'air de nous raconter une histoire où il y a plus que l'ingérence puisque des des des articles n'ont pas été produit sur. Sur injonction ou en tous les cas, les auto-censure très forte. Donc cette question-là moi à vise pas le service public je pense pas que c'est dans le service public qu'il y a. Ah. Un vrai sujet d'impartialité, d'informations, je pense que les processus de fabrication de l'information. La déontologie, la qualité des journalistes. La tradition de cette maison c'est que. La maison autant à Radio France, d'ailleurs qu'à France Télévisions. Faut que, à mon avis c'est probablement là où ça existe le moins Je pense que globalement dans tous les conseils d'administration des grands groupes qu'il soit privé au public. Un tel administrateurs peut être une bonne sentinelle. merci donc. Amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. pour. Est contre. Qui s'abstient et adopté. Nous passons à l'amendement suivant le 30, madame Robert. auront toujours le titre de président afin de garantir une certaine autonomie aux sociétés englobées sous cette Holding n'est pas opportun de faire de leurs dirigeants de simples directeurs généraux notre amendement tend donc à transformer ces directeurs généraux en présidents directeurs généraux. Loin d'être un simple symbole cette appellation ouvrira surtout le droit aux dirigeants concernés de présider leur conseil d'administration et non pas seulement d'assister le PDG de France Médias. Merci monsieur le président. Il est très important que le président directeur général de la société Holding soient également président non exécutif du conseil d'administration des quatres filiale pour veiller à la cohérence de la mise en oeuvre de la stratégie commune. À noter cependant que l'alinéa 23 de l'article 3 prévoit que les directeurs généraux seront par dérogation à l'article 93 tiré de de la loi du 29 juillet 1982, directeur de la publication. Ils conserveront donc la responsabilité entière de la ligne éditoriale. La Holding doit se limiter à la définition de la stratégie et à la répartition des moyens, c'est un avis défavorable. Sur le président avis défavorable également. Bien, donc un double avis défavorable sur cet amendement, je le soumets aux voix qui est pour. Qui contre. Qui s'abstient n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement suivant avec un sous-amendement mais l'amendement est présenté par. Monsieur Hugonnet. La commission. Merci, monsieur le Président, tenant compte des avis et du travail qui a été fait depuis cet amendement vise à simplifier le processus de sélection du président de France Médias et à renforcer les garanties concernant le choix des candidats. La nomination par décret en conseil des ministres est abandonnée au bénéfice d'une nomination par l'Arcom. Toutefois, c'est le conseil d'administration de la société qui aura la responsabilité de proposer un nom à l'Arcom comme il lui revenait de proposer un nom au président de la République afin de renforcer les garanties attachées au processus de sélection. L'amendement prévoit également la création d'un comité de nominations au sein du conseil d'administration qui devra veiller à garantir la transparence des critères de sélection, l'équité entre les candidats et la compétence des personnes dont il soumet le les noms au conseil d'administration, le comité de nomination aura l'obligation de soumettre au moins de nom au conseil d'administration de même c'est l'Arcom qui aura le pouvoir de retirer son mandat au président de France Médias et non plus le chef de l'État toujours suite à une décision motivée du conseil d'administration. pour que tout le monde comprenne. Nous avions proposé un amendement qui revenait à une nomination par l'Arcom. Le rapporteur en sortant cet amendement et je suis content qu'il ait été. Fait tomber le nôtre mais dans le note il y avait un 2ème élément qui me semble important. Par rapport à à l'expérience que l'on a connu. En gros moi la grande satisfaction que j'ai pu avoir pour avoir participé à la. de la loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. C'est que certes, c'était l'Arcom qui nommé. Mais il y avait eu énormément de plaintes et de doute porté. Sur la façon dont on ça avait été fait parce que il n'y avait pas eu publicité des débats. Et donc, ce manque de transparence laisser libre cours à une remise en cause. À un doute à une suspicion qui étaient jeté sur l'art comme probablement. Infondées, mais en tous les cas, je m'étais dit pourquoi on a oublié de traiter cette question de la transparence qui dans tous les processus aujourd'hui de délibération et de très important pour nos concitoyens, très important pour la démocratie. Donc ce que je propose que nous proposons c'est. D'ajouter cet élément qui existaient dans notre amendement mais qui n'existe pas dans celui de Monsieur Bonnet, c'est que pour la dernière phase. De nomination donc pas pour les La multitude des candidatures au début mais pour celles qui sont retenus dans la short list, il puisse y avoir. Des auditions en Direct et ouvert comme on le fait pour Public Sénat et le choix ici c'est comme ça que c'est fait pourquoi on le ferait pas J'ai entendu les arguments je je je l'ai développerait en ensuite parce que j'ai pu avoir le temps du rapporteur en commission, il a dit. Si les gens se manifestent et sont connus. Alors il ne candidate pas parce qu'ils abandonnent des postes importants, et donc, personne ne vient du privé candidatait. Et donc ça, c'est ce qui renforce l'opacité. C'est-à-dire que cette idée que il ne faut pas qu'on sache qu'on est candidat, si on n'est pas sûr d'avoir gagné, parce qu'on va abandonner son poste. Ça c'est pas possible dans le temps cet argument je développerai pourquoi tout à l'heure. C'est la transparence qui doit régner. Et c'est cela qui renforcera. L'indépendance de la décision, son autorité, sa crédibilité. Merci cher collègue alors. Donc l'avis du rapporteur sur le sous-amendement. Merci, monsieur le Président c'est ce sous-amendement n'a pas pu être. Vu tout à l'heure par la Commission puisqu'il arrive en séance. Donc c'est un avis personnel que je donnerai qui est un avis défavorable.

D'accord. C'est ce qui a été transformé en sous-amendement peut-être que j'ai noté. Mon. L'amendement 28.

Donc, cet amendement est primordiale. Je suis heureux qu'un autre amendement propositionnelle de dernière minute de notre rapporteur rejoignent en partie seulement nos préoccupations. Nous ne sommes donc pas les seuls hein. Satisfait de la proposition de nomination par décret. Telle que je le disais dans le la DG sur proposition du CA avec avis conforme de l'Arcom éventuellement véto. Des 3 cinquièmes des membres des commissions compétentes du Parlement. Nous souhaitons prévoit la nomination par l'Arcom du président directeur général de France Médias comme actuellement, mais nous entourant le processus de nomination de davantage de transparence par une plus grande publicité sur les candidatures des projets et les auditions des candidats. J'ai entendu l'avis de notre rapporteur sur cette question en commission qui estime que la publicité existant actuellement autour des candidatures empêche toute candidature d'une personne employée par le secteur privé, au risque de nuire à sa carrière en cas de rejet de sa candidature et si celle-ci venait à être connu. Je ne partage pas cette façon de penser. Je pense qu'une expérience préalable ou le secteur audiovisuel public comme dirigeant journaliste constitue une expérience appréciable et un plus non négligeable permettant d'être au fait des atouts et des arcanes du secteur. Il existe des précédents de candidats. Nommé à la présidence d'une société de l'audiovisuel public arrivant du secteur privé. Je me souviens de Jean-Pierre Elkabbach. Nommé en 93 par le CSA à la tête de France Télévisions, ils venaient d'Europe 1. Nous vous renvoyons au décret le soin de préciser les modalités de publicité des auditions des candidats parce que bien entendu, c'est quelque chose qui doit être très organisé. Comme indiqué dans l'objet de l'amendement. Nous ne souhaitons pas la publicité de l'ensemble des auditions de l'Arcom. Nous pensons qu'il serait opportun de rendre public seulement la dernière phase des auditions, celle des candidats de la short list afin de ne pas un influencer les unes les autres du fait de cette publicité des auditions les candidats pourraient par exemple être convoqués simultanément être auditionné dans un an de passage déterminé par tirage au sort, mais ça c'est le décret qui pourra le préciser je je je le répète ne sous-estimez pas. je dirais dans l'explication de vote. La réponse à à monsieur Gonnet. Donc, donnez votre avis monsieur le rapporteur, sur l'amendement 28 et puis ensuite. La ministre s'exprimera sur les trois. Merci monsieur le président la vie avait déjà été donnés en commission sur le 28, c'est un avis défavorable et pour la bonne et simple raison c'est qu'il les jumeaux du sous-amendements. Défavorable de la commission sur le sous-amendement et l'amendement qui suit, Madame la Ministre sur les trois l'amendement du rapporteur et les les autres. Merci monsieur le président. Sur le principe je salue cette modification puisque. Ça permet effectivement plus d'indépendance par rapport à la rédaction initiale, mais finalement ça revient à la situation actuelle, si on imagine qu'il n'y aura pas de Holding avec la nomination actuelle par l'Arcom des dirigeants. C'est donc la bonne garantie de l'indépendance sur ça je suis évidemment d'accord mais étant donné que je ne suis pas favorable, que le gouvernement n'est pas favorable, la création de la Holding je serai défavorable à l'amendement et sous-amendements merci. Alors nous avons donc un avis bon là le rapporteur et évidemment pour son amendement un avis défavorable sur l'autre et un avis défavorable pour l'ensemble de la ministre. Monsieur Assouline. je veux vraiment qu'on prenne la mesure. Bien entendu, nous sommes contents Holding donc tout ça c'est c'est des amendements qu'on appelle d'appel. De débat puisqu'on nous invite ici à un débat. Et donc je je veux pointer quelque chose. Qui a été très important qui est un manque. Même dans le système actuel. Quand il y a une délibération de l'Arcom de ce type. Il y a à chaque fois. Des suspicions sur la façon dont la délibération, c'est fait. Alors certains dit il y a eu des pressions d'autres il y a eu des. Des candidats plus ou moins défavorisés. Il y a eu. Des du favoritisme et etc. Et ça, il y a aucune maîtrise. De ce genre de rumeurs. Des fois ça pourrait être vrai. Pourquoi pas mais ça peut être fou en tous les cas ça entache la nomination. De. D'une opprobe J'insiste, si on veut encore parfaire le système des domination actuelle hein là c'est l'occasion du débat sur. Sur quelque chose qui n'existera pas probablement mais c'est pour le mode d'aujourd'hui que je pars. Il faut absolument réfléchir à la transparence de la délibération que chacun soit juge de la qualité des projets et de du foie et des raisons du choix que finalement l'Arcom. A fait. Merci donc. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Mais je souhaite prendre la parole à à cet instant parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les faiblesses de l'audiovisuel public demeurent nombreux aujourd'hui. On peut être d'avis diverses mais le développement numérique limiter la création audiovisuelle. Peu original et inadapté à l'exportation, l'offre d'information en continu déséquilibré entre radio, télévision et télévision offre de proximité peu cohérente et non coordonnées, la responsabilité de cette situation est partagé la tutelle n'ayant pas de compétences particulières en matière de stratégie de développement des médias, il ne lui a pas été possible au cours des 10 dernières années de définir une feuille de route claire. Mais les modalités de nomination des présidents par le Faute de pouvoir garantir la confidentialité des candidatures non pas non plus permis de choisir les personnalités, les mieux à même d'engager ces transformations aussi rapidement et profondément que nécessaire. Le nouveau mode de nomination qui est proposé. Par la Commission Ali le professionnalisme des mode de nomination des grandes entreprises à l'indépendance de l'Arcom cette procédure nouvelle pourrait permettre de trouver enfin un compromis acceptable par tous, permettant de conforter le professionnalisme et l'indépendance de l'audiovisuel public.

Qui s'abstient. Il n'est pas adopté donc nous passons maintenant à l'amendement de monsieur Hugonnet qui est pour cet amendement. Qui est contre.

Inutile de rappeler que c'est un amendement de repli. Bien entendu qu'il ne vient pas. Nous faire accepter ou quoi que ce soit la Holding mais de participer à ce débat, par les moyens qui. Qui nous sont données cet amendement de repli a pour objet de maintenir le même niveau d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du président directeur général que celui dont il dispose légalement aujourd'hui sur celle des présidents des sociétés de l'audiovisuel public notre amendement reproduit donc le dispositif malencontreusement oublié dans la rédaction de la PPL permettant d'assurer l'information du Parlement et son contrôle sur l'action des présidents de chaînes publiques de Radio France et de l'INA. Mais en l'adaptant quelques. Pour plus d'efficacité. Je suis très surpris que le Sénat redonne la main à l'exécutif sur la question du service public audiovisuel et se dessaisissent de ses pouvoirs de contrôle qui ne sont pourtant pas excessif. Ah. Ainsi notre amendement prévoit que 6 mois avant la fin du mandat du PDG de France Médias. Soit un an avant son terme l'Arcom rendra un avis motivé sur les résultats de la société France Médias au regard de son projet stratégique et de la réalisation de la convention. Avis qui sera transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, la commission chargée de la culture pour organiser une audition du président sur cette base. Par ailleurs, 2 mois après le début de son mandat, le PDG transmettra aux commissions de la culture de ces mêmes assemblées son rapport d'orientation et celles-ci pourront l'auditionner sur cette base, je ne pense pas trahir de secret en affirmant à quel point les auditions que nous menons sur ces bases de tiennent à coeur. Il s'agit d'un moment solennel est davantage qu'une formalité inutile, nous si on pas ne s'y ont pas nous-mêmes la branche sur laquelle nous sommes assis et maintenant les droits du Parlement, et notamment celui de contrôle de l'action des dirigeants ou du dirigeant de l'audiovisuel public. Merci monsieur Assouline. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Cet amendement prévoit les modalités d'information du Parlement concernant le projet stratégique du président de France Médias au début de son mandat et le bilan de son action au terme de son mandat. Ces dispositions qui figurait dans la loi du 30 septembre 86 apparaisse utile au regard de leurs objectifs la rédaction retenue permet par ailleurs d'obliger le président de la Holding à rendre compte régulièrement de son action devant le Parlement, ce qui est effectivement une bonne chose. C'est un avis favorable. Madame la Ministre. Monsieur le président. Sur le principe je suis toujours évidemment favorable à ce que le Parlement puisse être. Le mieux informé possible mais vous avez déjà la possibilité d'auditionner à tout moment les entreprises l'Arcom. Les rapports existent son public. Pour ma part, ce serait un une demande de retrait. Qui est contre. Il s'abstient. Il est pas adopté amendements suivant le 55 rectifié madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement reprend la 2ème partie de la proposition numéro 26. Qui avait été adopté à l'unanimité des membres de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias tout à l'heure, nous avons voté la mise en place d'un administrateur indépendant chargé de veiller à l'impartialité de l'information dans les sociétés de l'audiovisuel public. Cette proposition préconisait de cet administrateur rende compte annuellement de cette impartialité devant les commissions chargées des affaires culturelles et des médias, des 2 assemblées tel logeait de cet amendement qui prévoit donc cette information au moment où les commissions le jugeront opportun.

l'impartialité de l'information du service public, constitue une impérieuse nécessité pour assurer la légitimité du service public. Le fait que le Parlement puisse interroger celui qui aurait la responsabilité de défendre ce principe répond également à une nécessité, c'est un avis favorable. Madame la Ministre. Même avis par rapport à ce que j'ai dit précédemment, l'impartialité, c'est vraiment un sujet très important pour l'audiovisuel public comme privé. Mais en cohérence avec mes positions précédentes. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. donc un avis favorable de la commission demande de retrait ou avis défavorable du gouvernement. L'amendement est maintenu, j'imagine. Donc, je le soumets aux voix qui est pour.

Il s'abstient. Il est adopté. Nous passons aux amendements sur l'article IV avec quatre amendements identiques de suppression monsieur Bargeton. Défendu. Monsieur Assouline. Défendu monsieur. S'est fendu. Madame de Marco. Non je le défends. L'article 4 est un simple amendement de coordination qui s'inscrit dans le même objectif de constitution d'une Holding chapeautant les sociétés audiovisuelles publiques. Le projet de directive européenne sur la liberté des médias qui a été présenté par la Commission européenne en septembre dernier prévoit des règles et mécanismes pour un financement adéquat de sable et transparent des médias de service public. Nous devrions anticiper. L'entrée en vigueur de cette directive plutôt que de perdre du temps à légiférer sur des dispositions contraires à cette directive européenne. Merci à vie de monsieur le rapporteur. Sur ces quatre amendements de suppression. Ce sont 4 amendements de suppression. Monsieur le Président, c'est donc un avis défavorable. Merci, madame la Ministre. Avis favorable aux suppressions. Qui est contre. Qui s'abstient. L'article 4 est adopté. Nous passons aux amendements de l'article 5. Avec 3 amendements identiques de suppression.

remercie Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. L'audiovisuel extérieur est un outil essentiel au rayonnement culturel de la France en soutien à la francophonie, c'est également un atout puissant pour porter notre parole est diffusé notre vision du monde sur une scène internationale dominée par les médias anglo-saxons malheureusement ce texte qui propose principalement la création d'une Holding chapeautant les 3 sociétés de diffusions publiques de l'audiovisuel. France Télévisions, Radio France Radio France et France Médias Monde ainsi que l'INA ne ferait qu'affaiblir cet outil dont je viens de démontrer l'importance comme l'a évoqué mon collègue David Assouline, cette volonté de rassemblement de 4 sociétés dont les missions et public sont très différents. Risque d'engendrer une uniforme et Asia sur des programmes qui nuirait à leur diversité et pourraient ne plus répondre aux fortes attentes notamment des communautés francophones et francophiles dans le monde. Par ailleurs, vous proposez que cette Holding et les mains libres pour répartir les ressources qui lui seront attribués entre ces sociétés. Le Parlement ne sauraient qu'informé de cette répartition alors qu'ils contrôlent aujourd'hui les dotations. Monde qui comprennent qui comprend notamment, France 24 et RFI et dont le chiffre d'affaires est bien inférieur aux autres risque fort d'être mis en minorité à la table des négociations et ainsi de faire les frais des ajustements budgétaires nos compatriotes établis hors de France. Ils sont pourtant très attachés. TV5 Monde et Arte qui n'entre pas dans le dispositif. Le premier parce que son capital n'est pas intégralement détenu par l'État. La seconde parce qu'elle est régie par un traité bilatéral risque elle aussi d'être mise à l'écart. Je crains que l'audiovisuel public extérieur ne soit pas la priorité pour ne pas dire le grand perdant de cette proposition de loi. Et pour toutes les raisons évoquées par mon groupe auquel j'ajoute ces lacunes. Je voterai contre ce texte, à un moment où je voudrais ajouter quand même que la désinformation et la propagande organisée par certains États nous force à avoir une parole qui soit entendu, écouté à l'étranger. Merci.

qui a. Été jugée recevable. Article 40 donc j'en profite pour en parler sinon j'en aurai pas l'occasion. Ce dernier c'était un amendement de repli qui reprend l'une des dispositions contenues dans la proposition de loi de notre groupe qui visait à assurer la qualité d'indépendance du service public de l'audiovisuel par un financement affecté juste et pérenne. Il tend à modifier la loi du 30 septembre 86 relative à la liberté de communication afin de graver dans ce texte le principe d'une ressource dédié aux sociétés de l'audiovisuel public provenant d'un nouveau front de contribution progressive à l'audiovisuel public. Alimenté. Par une contribution annuelle universelle et progressive versés par tous les ménages non dégrevés de cette contribution. La création d'un fonds dédié à l'audiovisuel public graver dans la loi de 86 serait complété par le contrôle annuel par une commission indépendante du montant et de la répartition des sommes destinées à l'audiovisuel public. Cette commission serait composée de 2 sénateurs de députés de représentants des usagers et présidée par un haut magistrat de la Cour des comptes elle aurait la faculté de s'auto-saisir cette garantie de contrôle indépendant sont est d'autant plus nécessaire que le gouvernement français au lieu de moderniser la redevance, à l'instar de ce qui a cours chez nos voisins européens a créé un précédent en revenant sur le caractère pérenne et infecté de la ressource dédié à l'audiovisuel public pourtant garante de son indépendance et donc du pluralisme et de la démocratie. Au sein des médias, je tenais à pouvoir le dire. Autrement que par un amendement. Et voilà pourquoi j'ai demandé une parole. donc. Après ces 2 interventions sur article nous reprenons l'examen des amendements donc je disais qu'il a sur cet article. Trois amendements identiques de suppression. Le premier de modules Bargeton défendu. Le seconde monsieur Assouline. Défendu amendement de suppression. Oui sur le cinq. C'est madame Robert. Le 16. Oui le 16. Merci monsieur le président, bien cet amendement tend à supprimer l'un des articles phares concernant la Holding. Puisque c'est celui qui institut les futures conventions stratégique pluriannuel ainsi que les modalités d'information et de suivi du Parlement et enfin le dispositif qui prévoit le mode de financement du service public de l'audiovisuel. Film garantit que certains au sein de cette assemblée. Ne semble même pas vouloir assurer si j'en crois le dépôt de l'amendement de suppression de l'alinéa concernés. Ces conventions stratégique pluriannuel qui remplaceront les actuels comme auront une durée maximale de 5 ans et aucune durée minimale, alors que les comme avaient une durée de 3 à Pourquoi ne pas garder une durée minimale, alors que l'on déplore fréquemment la stabilité des dotations budgétaires En outre, ces conventions pourront-ils caduc et renégocier en cas de l'arrivée d'un nouveau président, ce sera donc une instabilité qui pourraient être préjudiciables contrairement aux actuels comme ses futures convention n'auront plus à comporter d'engagements en matière de création d'information de diversité. La PPL ne leur donne comme objectif que ceux de gestion et de comptabilité. La vocation informative éducative, culturelle et de divertissement du secteur public de la vie de l'audiovisuel semble donc être très accessoire tout comme bien sûr son accessibilité à différents publics. La preuve est donc faite que le projet de la majorité sénatoriale pour l'audiovisuel public est un projet contre celui-ci. Le seul objectif étant un resserrement de son financement afin que les marchés profitent au mieux des services audiovisuels privés et au développement de la recette. Merci et ensuite l'amendement en 89. Madame de Marco. Merci. L'article 5 propose de remplacer les actuelles conventions d'objectifs de moyens. Par des conventions stratégique pluriannuel établi entre l'État et les sociétés. Public, nous y sommes opposés parce que nous sommes opposés au projet de Holding défendue par l'auteur de la proposition de loi. Nous avions proposé un amendement visant à améliorer le fonctionnement des contrats d'objectifs et de moyens afin de renforcer l'indépendance de l'audiovisuel public et d'améliorer leur visibilité budgétaire. Comme le souligne le rapport de l'IGA assez et de l'IGF de 2022 relatif au financement de l'audiovisuel public sur la période 2011 2022, les engagements financiers des comme ont été sans cesse réécrit. La plupart du temps les engagements pris par l'État n'ont pas été respectés. C'est pourquoi il était proposé d'exclure la possibilité de procéder à des avenants modifiant à la baisse des ressources allouées. Il ne me semble pas que cela constitue une aggravation des choses publiques. Mais la commission des finances un a décidé autrement. Enfin. Afin de garantir l'indépendance du pouvoir public nous proposions de porter la durée des comme à six ans afin d'améliorer la visibilité mais aussi de décoller. Décorrélés le temps des comme des cycles électoraux électoraux en application des des recommandations européennes. Merci. Avis du rapporteur sur ces trois amendements de suppression. Merci monsieur le président. Sans surprise, comme ce sont des amendements de suppression et qu'il supprime un élément important du dispositif, c'est un avis défavorable sur les trois.

que le prochain contrat d'objectivité de moyens soit de 5 ans pour justement enjamber. La, la période des élections futures puisque ça va être de 2024 à 2028 après une prolongation d'un an des contrats d'objectifs et de moyens actuels. Et j'en profite. Ce que tout à l'heure monsieur le rapporteur. Vous avez dit que la création audiovisuelle n'était pas adapté à l'exportation et on n'a pas encore parler de l'impact international des des productions. Là tout de même, je trouve que il y a. Un véritable succès pour les productions de France Télévisions. Regardez le succès mondial de 10%. Regardez le nombre de pays qui ont décliné Fort Boyard les coproductions, le tour du monde en 80 jours Germinal Léonard de Vinci. La nouvelle série abysses. Coproduite avec l'Allemagne, l'Italie qui a un démarrage très fort l'animation aussi qu'ils ont très bien à l'international. Je vais me rendre jeudi à Annecy pour le festival d'animation et France Télévisions est un des principaux financeurs de l'animation française donc là honnêtement je trouve que votre constat est un peu sévère. En tout cas. Avis favorable aux suppressions. donc un avis défavorable du rapporteur sur ces amendements de suppression un avis favorable du gouvernement. Je les soumets on voit donc il est pour les amendements de suppression. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés

Cet amendement tend à fixer une durée minimale aux futures convention stratégique pluriannuel. La proposition de loi ne fixe que la durée maximale qui restera de cinq ans comme celle des actuels les sociétés pour mener à bien leur projet ont besoin de stabilité et ne pas se voir modifier leur convention tous les ans voire au bout de quelques mois, ce qui serait possible en vertu du dispositif proposé sans durée minimale. Je m'étonne d'ailleurs d'une maintien des actuels comme dans leur périmètre alors qu'ils sont en cours de renégociation entre le gouvernement et les sociétés concernées. Quel est le but de cette modification mise à part celui d'un cadre moins disant sur le plan qualitatif ou des garanties. On a assez déploré de les nombreux avenant au COM intervenues ces dernières années, dont le seul but était de rogner les financements du secteur public audiovisuel sous le couvert d'un plan d'économies de près de 200 millions en 5 ans, il n'est donc pas opportun que la loi fragilise encore davantage le dispositif l'amendement proposant de fixer une durée minimale légale aux conventions et de la maintenir à trois ans durée correspondant à celles prévues pour les comme actuel. Et avis du rapporteur. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à prévoir que la convention stratégique pluriannuel ne pourra pas avoir une durée inférieure à 3 ans afin de favoriser la stabilité des sociétés France Médias et de ses filiales et d'Arte France. L'objectif de stabilité très important et on peut effectivement s'interroger sur l'intérêt d'une convention stratégique pluriannuel dont la durée serait limitée à 2 ans. D'autant plus que la rédaction de l'article 53 prévoit déjà la possibilité de conclure une nouvelle convention après la nomination d'un nouveau président il n'est pas inutile de rappeler par ailleurs que le comme d'Arte France est subordonnée au contrat de groupe d'Arte GEIE dont la durée est habituellement de 4 ans, c'est donc un avis favorable. Madame la Ministre. Monsieur le président. J'ai déjà indiqué ma position sur le besoin de visibilité pour les entreprises d'où les contrats d'objectifs et de moyens proposés pour 5 ans mais par cohérence avec mes positions. Défavorables à la Holding. Je suis défavorable. Bien je soumets l'amendement voit avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui pourront. Qui est contre. Il s'abstient. Il est adopté. L'amendement 32 de monsieur Assouline. Merci monsieur le président. Cet amendement tend à éviter un facteur d'instabilité supplémentaire au secteur de l'audiovisuel public. N'est pas opportun effectivement de fragiliser davantage ces sociétés en prévoyant une possibilité de renégociation de la convention stratégique pluriannuel en cas de changement de président. Cette possibilité, pourrait notamment permettre de renégocier à la baisse les financements de la société. Or on le sait, l'audiovisuel public a besoin de stabilité pour mener à bien ses projets en poussant le raisonnement à l'extrême, on pourrait même imaginer que le dispositif pourrait inciter un changement de président, afin de pouvoir modifier une convention. Pourquoi pas et même rogné les financements de de cette société. Il s'agit donc, pour nous d'une disposition très dangereuse et nous en demandons la suppression je profite de cet amendement pour regretter une fois de plus les recevabilité au titre de l'article 40 de notre amendement 36 car non compatible avec les termes de la LOLF. Nous souhaitons en effet l'annexion des conventions au projet de programmation pluriannuelle des finances publiques, ce qui les aurait lié au vote de cette programmation l'état se trouvant alors davantage en gaz et je suis sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public. Le Parlement ne se prononcera plus sur la répartition de la ressource publique entre les sociétés c'est très partition ne figurera plus dans les projets annuels de performances budgétaires qui ne fera apparaître que la dotation globale. globale. À France Médias. Ce manque de transparence est inacceptable pour les législateurs que nous sommes contraire à la règle d'annualité budgétaire que le son conseil constitutionnel a érigé en principe constitutionnel et dangereux pour le maintien de de l'audiovisuel public dans son périmètre actuel. Merci, madame Robert. Avis du rapporteur sur cet amendement. autant il n'apparaît pas judicieux de supprimer de la possibilité d'adopter une nouvelle convention en cas de changement de président le rôle du président et d'élaborer la stratégie de la société et il n'apparaît pas opportun d'obliger un nouveau président à mettre en oeuvre les priorités de son prédécesseur. C'est un avis défavorable. Avis défavorable. Madame la ministre. Même avis que le rapporteur. Donc un double avis défavorable sur cet amendement. Qui est pour. L'amendement. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 33. Madame Conway Mouret. Merci Monsieur, Monsieur le Président, vous souhaitez que les conventions stratégique pluriannuel soit moins disante. Sur le plan culturel que les actuels comme avec aucun engagement en faveur de la création ou de l'information. Nous vous l'avons d'ailleurs déjà fait remarquer. Nous voulons au contraire que ces conventions soient plus ambitieuses pour que le service public audiovisuel joue le rôle qui doit être le sien en faveur de la création et du soutien aux industries culturelles. Il doit continuer à être un moteur et à financer des productions et coproductions ambitieuse. Le monde du cinéma et de la production audiovisuelle connaissent leurs besoins de financement. Et d'exposition de leurs Oeuvres pour les prochaines années nous semblerait donc pertinent d'associer leurs représentants à la négociation des conventions. Cet amendement a pour objet de préparer la négociation et la rédaction des conventions stratégique pluriannuel dans une des plus grande transparence et dans un but de meilleure adéquation avec les objectifs et réalité des milieux de l'information et de la création. Une fois n'est pas coutume, ça t'amendement rejoint les. Occupation exprimée par la Commission bataillon et sa proposition numéro 27. Merci. Merci monsieur le président. La vie sur cet amendement 33 le remplacement des comme par des conventions stratégique pluriannuel vise à simplifier ces documents et rentrent dans leur préparation plus simple pour les sociétés. L'État et le régulateur si des consultations sont bien évidemment souhaitable le présent amendement ne précise pas qui serait chargé de les organiser à quel moment et pendant combien de temps. C'est peut être le rôle ce peut être pardon le rôle du Parlement de concourir à ces consultations dans des formes propres au travail parlementaire. C'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur. Si je me place dans la situation actuelle. Comment les contrats d'objectifs et de moyens sont en train d'être préparés, ça fait plusieurs mois que ces concertations ont lieu je vous et, vous-même, invitée d'ailleurs à plusieurs réunions, nous avons fait un certain nombre de de consultations, il y a eu énormément d'audition également à l'Assemblée comme au Sénat. Donc ça existe déjà. En tout cas même avis que le rapporteur.

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, je suis plus que surpris de l'absence de projet ambitieux de ce texte pour le secteur audiovisuel public dont les seuls objectifs selon le dispositif serait à l'avenir budgétaire et comptable. Ce n'est pas sérieux. Les comme actuels ont sans doute des défauts, mais la loi les encadre de façon à permettre la contribution des sociétés de l'audiovisuel public, à l'industrie de programmes au développement d'une information de qualité au maintien de la culture française à l'accessibilité des programmes à tous les publics, dont ceux souffrant de handicap. Votre amendement ton donc intégré dans les mentions devant figurer dans la future convention stratégique pluriannuel celle devant aujourd'hui figurer dans les comme. Nous reprenons donc simplement la rédaction actuelle de l'article 53 afin de garantir dans ces conventions la vocation informative éducative, culturelle et de divertissement en direction de tous les publics du secteur public de l'audiovisuel en l'état cette PPL aura pour conséquence d'appauvrir l'industrie de programmes de faire reculer la francophonie et d'isoler les publics souffrant de Andy. puisque ces références ne sont plus mentionnés pour laisser la place aux chiffres et à la comptabilité, un projet de Holding. De cette sorte. Mais franchement pas à visage humain. Merci. pluriannuel pardon vise précisément à éviter de multiplier les thèmes abordés ce qui aurait inévitablement pour conséquence de transformer ces documents catalogue de bonnes intentions sans véritable portée opérationnelle comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci, monsieur le Président, c'est également un avis défavorable. Même si sur le fond je comprend complètement que vous souhaitiez réaffirmer ses enjeux en réalité sont déjà dans la loi de 86, les 2. Engagements que vous voulez insérer. Après l'alinéa 4 les engagements anti-de la diversité de l'innovation dans la création les montants minimum d'investissement c'est déjà dans la loi de 86, ces principes là. Quant aux engagements. En matière. De d'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est dans le cahier des charges, en réalité c'est ça existe des gens avis défavorable. Bien, donc un double avis défavorable sur cet amendement je me soumets on voit qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Donc maintenant nous avons 3 amendements de suppression de l'alinéa 10 de cet article 5. Le premier, le 35 monsieur Assouline.

Pour le service public mais qui pourrait se révéler assez fructueuse pour les services audiovisuels privés. Elle a été introduite en commission sur proposition du rapporteur qui sous couvert de je cite mieux distinguer et préserver l'offre de service public a prévu que la convention stratégique pluriannuel fixera le les recettes commerciales donc publicité parrainage des différentes sociétés en fonction du niveau de ressources publiques prévues. Le budget global des sociétés serait ainsi gelée et plafonné pour plusieurs années. Dès la rédaction de ces conventions et sans sans avoir et ce pardon sans avoir connaissance des aléas pouvant affecter l'économie pendant la durée de la convention. En vertu de ce dispositif. Seules les sociétés privées l'audiovisuel pourrait profiter d'un marché publicitaire soudainement en bonne santé et non les sociétés publiques malheureusement tenu par les conventions plafonnant leur budget global et restreignant leurs objectifs commerciaux. Donc voilà l'objet de cet amendement. Monsieur le président. Merci. Monsieur Bach Merci Monsieur le Président. Nous sommes favorables à un haut de audiovisuel public sans publicité et ça pourrait tout à fait être une différence notable avec les acteurs privés il faut financer l'audiovisuel public, trouver d'autres. Sources, d'autres recettes que ne prévoit absolument pas le texte qui nous occupe aujourd'hui, on a déjà l'expérience de l'arrêt de la publicité après 20h qui devait être compensée et qui ne l'est finalement plus. Et cette proposition de loi qui prétend vouloir armer l'audiovisuel public face aux plateformes et aux acteurs privés. Qui dispose de moyens considérables, on le sait finalement des armes, l'audiovisuel public. Tout en lui demandant de développer de nouvelles offres. On a évoqué notamment le numérique. Mais non, non content de désarmer le secteur public. Elle renforce la concurrence déloyale avec le privé puisque les plateformes et l'ensemble des acteurs privés. Bénéficieront de ses recettes publicitaires qui ne n'iront plus vers l'audiovisuel public et donc on est là dans, dans deux dispositions est extrêmement dangereux effectivement pour l'audiovisuel public, qui a besoin de moyens conséquents face. Aux autres acteurs qui lui mène une concurrence redoutable.

Mais l'article 5 relatif aux conventions stratégique pluriannuel a été amendé en commission par le rapporteur. Et il a rajouté la mention selon laquelle les recettes publicitaires et de parrainage devraient être plafonné par la dite convention. on vit, on vient plafonné je le budget, l'audiovisuel public, déjà fortement contraint. Alors qu'on a déjà adopté la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Mais comme si cela ne suffisait pas. Comme ce n'était pas suffisant de brider les ressources du public. Le rapporteur a aussi fait adopter un amendement autorisant les chaînes privées à réaliser jusqu'à trois coupures publicitaires par film diffusé d'un côté pour le public on limite on plafonne. De l'autre pour le privé, ont dérégulé, on laisse faire, il y a 2 poids 2 mesures assez révoltant c'est assez hypocrite quand on regarde le texte dans sa globalité. Évidemment je ne souhaite naturellement pas l'une extension de la publicité dans quelques médias, que ce soit mes engagements sur d'autres textes sont constants. Ce que je souhaite en revanche c'est qu'au lieu de corseter les revenus. La télévision publique notamment issus de la publicité, on s'interroge, d'abord sur la manière de créer des des financements suffisant et durable. Supprimer la publicité oui 1000 fois oui mais pas avant d'avoir trouvé des financements durables et surtout pas si l'on impose des règles au public en laissant prendre au privé la voie strictement inverse. Merci. Avis du rapporteur sur ces amendements de suppression. d'un plafond de recettes publicitaires et de parrainage apparaît indispensable pour mettre un terme à la dérive actuelle qui voit, France Télévisions et Radio France recourir de plus en plus à la publicité et au parrainage, faute d'être capable de rationaliser leurs dépenses et de faire des choix stratégiques. Cette dérive est dangereux autant que l'hypocrisie pour la spécificité du service public et fragilise l'ensemble du secteur et notamment les entreprises qui ne peuvent disposer de dotations publiques qui demeure considérable. À noter que le montant du plafond serait fixé dans la convention stratégique pluriannuel ce plafond pourrait être dans un 1er temps consister à geler le montant des recettes publicitaires en attendant de développer des ressources alternatives liées notamment aux revenus générés par les investissements dans la production. Pour ce qui est de France Télévision, c'est un avis défavorable pour les trois amendements. Monsieur le président. Avis favorable du gouvernement aux amendements de suppression. Si les recettes publicitaires sont une. Ressource d'appoint pour le service public, elle n'en reste pas moins indispensable à son équilibre économique à l'accomplissement de ses missions. Et en réalité on a pu le voir en 2009. Quant la publicité après 20h a été supprimée, ce que les recettes qui ont été perdus par France Télévisions ne sont pas allés automatiquement vers les chaînes privées en réalité qui a capté le marché de la publicité depuis toutes ces années, ce sont les Gafam et continue à capter le marché de la publicité donc aujourd'hui le débat il est pour les chaînes privées comme publiques. La concurrence des Gafam, au fond c'est c'est ça le vrai sujet. En tout cas à plafonner les recettes publicitaires et de parrainage de France Télévisions pourrait au fond actuellement fragilisé la capacité de l'entreprise à à maintenir son niveau actuel de de soutien aussi à la création audiovisuelle et cinématographique française et mener à bien les investissements influe indispensable pour ses offres numériques qui doivent être renforcés. Donc, avis favorable aux suppressions. Bien merci donc un avis défavorable du. De la commission est favorable du gouvernement, monsieur Assouline. Oui c'est, c'est un débat important. Ou l'essentiel pour moi et et de faire sauter des des espèces de vérités assénées qui ne sont. Pourtant pas des vérités. D'abord, le marché de la publicité et du parrainage à France Télévisions ne représente que 1% du marché total de la publicité en France. Ces 3% du marché de la publicité TV et la pub digitale sur France TV c'est 04% du marché de la publicité digitale ont franchement c'est relativement marginal. Ensuite. Un élément important parce que là, il est culturel. Notre rapporteur monsieur Hugonnet. Nous dit. Oui. En gros la différenciation avec. TF1. Avec le privé se fait après 20h, par le fait justement qu'il y a pas de publicité. Or aujourd'hui, cette différenciation elle existe nettement parce que là où il y a 3 minutes il y a 40 minutes sur TF1 et de et donc ce n'est pas aujourd'hui le parrainage le volume du parrainage qui. Qui. Rend confus, le fait qu'on serait sur un TF1 bis je je je dis attention à, à ce qui est en train d'être fait parce qu'on nous l'a déjà fait. Sur la suppression d'après 20h. Le privé la réclamer. Le gouvernement l'avait fait, celui de Nicolas Sarkozy. Et puis finalement ça n'a pas été. Pour le privé ça été vers Internet et les Gafam que les compensations prévues à l'époque, hé bien n'ont pas été au rendez-vous puisque c'était la taxe. Sur. Les fournisseurs d'accès qui maintenant est captée entièrement par le gouvernement est pas reversé pour compenser pour France Télévisions, qu'on peut continuer à rogner, rogner et à aucun moment. Monsieur Bonnet vous prévoyez un dispositif de compensation. De cette recette. Ça veut dire que vous dites dorénavant qu'il y aura. Moins de recettes sur France Télévision. Je ne comprends pas et vous savez très bien aussi je veux finir là-dessus que quand on dit qu'il a un plafonnement pour une société qui va. Mais des personnels pour aller chercher la pub, c'est un travail si on le dit bah de toute façon, ne vous cassez pas trop la tête à aller chercher parce que si vous en faites trop, ça va être raboté parce que c'est plafonné. Hé bien on démobilise les équipes, on fait en sorte que même ce qui est accepté n'ait plus trouvé. Merci. Donc sur ces amendements. Nous donc. Procéder au vote Madame Morin-Desailly. Oui. Ce débat sur la publicité, on l'a longtemps eu au sein de cet hémicycle et je me souviens encore. Le, la proposition de loi qui a visé avec succès à supprimer la publicité. Sur les chaînes jeunesse de l'audiovisuel public. Il y avait une forte résistance de l'audiovisuel public. Vous pensez bien à supprimer ses recettes. Voilà pour cette chaîne particulièrement la jeunesse mais nous lui sommes arrivés car l'état d'esprit. C'est bien de différencier ce qui est le financement. Le modèle économique de diviser le public qui doit être libérée des contraintes commerciales et celui de l'audiovisuel public. Privé. Le vrai sujet pour moi, le vrai scandale, chers collègues, c'est la suppression pure et simple de la TOS, c'est-à-dire que, forcément, que l'audiovisuel public a eu tendance à accroître les parrainages et les tentatives de capter un peu de publicité ici et là, puisqu'au fur et à mesure des années, on n'a pas respecté l'engagement ce qu'avaient voté le législateur et je fais partie, comme David Assouline de ceux qui ont voté la toasts la création de cette taxe pour compenser la suppression de la publicité après 20h. Elle a cessé de diminuer depuis 2009 jusqu'à disparaître totalement il y a deux 3 ans, je me souviens plus tellement et la date exacte mais voilà où on en est là, donc le vrai sujet. Ça va être en loi de finances de savoir quelles ressources publiques et quelle compensation pour la suppression de la publicité après 20h, ni plus ni moins. Donc moi je voudrais connaître l'engagement de Madame la Ministre sur ce sujet de la tasse alors ça ne relevait pas de votre responsabilité Madame la Ministre que vous n'étiez pas ministre de la culture. Mais pourquoi a-t-on supprimé définitivement l'Athos et je trouve ça assez scandaleux qu'une taxe décidée par le législateur qui est une taxe affectée, avec un objectif précis soit complètement détourné de son objet et aille remplir le puits sans fond de Bercy point barre. Voilà ce qui est la réalité de la tasse aujourd'hui alors moi qui ai voté la tonne en 2009 en connaissance de cause ont supprimé la publicité après 20h sur France Télévision. Je ne suis pas très content de cette c'est aujourd'hui je vous le cache pas. Merci. Donc nous allons passer au vote, sur ces trois amendements avec un avis défavorable du rapporteur et un avis. Favorable de. La ministre qui est pour.

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir que la répartition des ressources publiques entre les sociétés sous tutelle de la Holding France Médias sera comme aujourd'hui débattu et voté lors de l'examen de la loi de finances annuelles. Afin de sécuriser les dotations de chacune des sociétés. Elle serait individualisé dans un fascicule dédié de projet annuel de performance présentée dans le cadre de la loi de finances. Je l'ai rappelé tout à l'heure ne défendant en défendant un autre amendement, d'annuaires d'annualité budgétaire a été érigé en principe par leur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel car découlant de l'article 47 de la Constitution qui dispose du vote de la loi de finances par le Parlement dans des conditions fixées par la LOLF. Par cette PPL, je le répète aussi nous allons renier nos pouvoirs et ce dans le seul but de faire plaisir à quelques acteurs du paysage audiovisuel privé et au détriment de l'intérêt du service public. Olivier. Audiovisuel et des téléspectateurs. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi notre rapporteur qui est parlementaire comme moi. Pensent qu'il est inutile de. Préserver le droit que nous avons aujourd'hui. De voter sur des montants pour chaque société de l'audiovisuel de les connaître, qu'il soit transparent de nous déposséder de ce pouvoir de contrôle. Je n'ai pas entendu de réponse je je lui demande vraiment de, de revenir à la dessus. Ce n'est qu'un amendement d'appel, de toute façon on sait très bien que que Holding. A peu de chances de voir le jour, mais en tous les cas, c'est pour ça que je suis un amendement de repli mais dans la logique même du rapporteur je ne comprends pas pourquoi il ne donne pas un avis favorable à cet amendement. Merci à Lille. Monsieur le rapporteur, justement. Merci, monsieur le Président, cet amendement reviendrait à remettre en cause tout simplement une compétence essentielle de la société Holding concernant la répartition des moyens en fonction des priorités. Il est très important que les priorités comme les moyens fassent l'objet d'une programmation dans le cadre de la convention stratégique pluriannuel et que les dirigeants conserve la souplesse nécessaire pour mettre en oeuvre ses priorités. Cette absence de souplesse et de capacité à définir des priorités est une des raisons principales des difficultés des sociétés de l'audiovisuel public, à l'heure actuelle, tout simplement, c'est un avis défavorable. C'est le président avis. Défavorable étant donné que je ne veux pas rentrer dans le débat de comment se réorganiser. Les dotations. Mais ce que vous venez dire monsieur le rapporteur, montre bien au fond que cette Holding va prendre énormément de place va nécessiter énormément de monde parce qu'il va falloir gérer. Tout le budget de tout l'audiovisuel public. Bon ça, ça ne va pas du tout être 20 ou 30 personnes, ça va être une énorme usine à gaz. C'est c'est juste ça que je perçois encore plus. Il y a un merci donc un double avis défavorable. Je soumets l'amendement voit qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement. 1er rectifié madame Estrosi Sassone. Oui, monsieur le Président très rapidement cet amendement qui est proposé par notre collègue Roger Karoutchi est co-signé par un certain nombre de nos collègues propose de supprimer la référence au financement des sociétés de l'audiovisuel public, telle que présentée à l'article 5. Merci monsieur le président et le financement de l'audiovisuel public constitue la principale garantie de son indépendance. Il est fondamental de défendre cette indépendance pour autant que celle-ci ne servira pas à maintenir des rigidités défendre des corporatismes et ralentir les évolutions indispensables. Dans notre esprit il est essentiel de réformer à la fois le financement, l'organisation et la gouvernance de l'audiovisuel public afin de mettre un terme à la situation actuelle qui mobilise des moyens considérables avec des résultats limités en particulier dans la capacité de ces entreprises à s'adresser aux jeunes à faire preuve d'innovation et d'originalité et à contribuer au rayonnement de la culture française à l'international. 2 scénarios sont dès lors envisageables. Un regroupement de l'audiovisuel public dirigé par une personnalité incontestable qui saura définir et mettre en oeuvre une stratégie ambitieuse avec des moyens suffisants. Ce scénario pourrait justifier d'allouer un financement pérenne et fiscales à la société Holding. Pourquoi pas en pérennisant le mode de financement actuel qui a fait ses preuves. Deuxièmement, le maintien de la situation actuelle caractérisée par un éparpillement des sociétés des structures trop coûteuse et assez pesé fit assez peu efficace des mutualisations cosmétique ce second scénario pourrait justifier de recourir à un financement par dotation budgétaire afin de limiter le coût de cet audiovisuel public le présent amendement anticipe l'échec de notre ambition pour un audiovisuel public moderne, dynamique et rénové. Nous ne pouvons qu'y être défavorable tant que l'issue de la présente, proposition de loi ne sera pas connu. Il faut se laisser une dernière chance. Cher collègue, avis défavorable. Sur le président. Avis défavorable à cet amendement qui supprime les caractéristiques. Du financement de le diésel public caractéristiques qui sont cohérentes avec les grands principes que j'ai réaffirmé à savoir que le que l'audiovisuel public bénéficie d'une ressource prévisible et suffisante pour lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont confiés et en tout état de cause, le débat sur le mode de financement pérenne du secteur va être défini en loi de finances, avis défavorable. Bien merci Madame Morin-Desailly. J'ai envie de dire, nous y voilà. La suppression de la redevance. C'était l'annonce de la re-budgétisation du financement de l'audiovisuel public. Notre groupe s'était opposé à la suppression à l'aveugle, l'été dernier de la redevance avait demandé une année d'études notamment ça émané de la, la commission de la des finances de nos collègues centriste de la commission des finances. Pour pouvoir d'abord bénéficié de l'étude de demander à l'IGAC car je vous rappelle chers collègues qu'on a dû quémander pour l'avoir et qu'on l'a eu en dernière minute. Donc pas de recul pour pouvoir fournir une solution satisfaisante assurant vraiment la pérennité et l'indépendance de l'audiovisuel. Public donc pour le moins, il était important que cette proposition de loi déposée par notre collègue Laurent Lafon comporte cette disposition qui affirme la nécessité d'une ressource pérenne dynamique. Lisible. Donc moi je soutiens absolument cet article maintenant il faut que ça se concrétise dans la loi de finances et que nous ayons des vrais débats sur ce qu'est la la ressource publique et je vous l'dit à cet égard à Madame la la Ministre que lors de la paix fut, il y avait un débat formidable organisé sur l'avenir de l'audiovisuel public en général avec les différents audiovisuel public européen qui sont venus et ils ont dit, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, pardonnez-moi de vous contredire Madame. Que la première condition de l'indépendance des entreprises de du Vidal public était bien le leur mort de leurs ressources et la ressource publique dont la contribution à l'audiovisuel public. Il a le mode de nomination. Mais il y a aussi la question de la ressource et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'en 2009 nous rebaptisant la redevance contribution à l'audiovisuel public. C'est pas une taxe, comme une autre, c'est une participation des citoyens à un financement dont ils bénéficient, avec des programmes qui leur sont dédiés des orchestres aussi qui sont financés grâce à cette ressource. Donc il y a une dimension citoyenne dans cette contribution sur lequel on aurait intérêt à débattre dans les temps à venir, en tout cas dans la perspective de la loi de finances, je vous remercie. Merci. Le président là font. mais très rapidement, on y vient à travers les nombreux amendements qui ont été déposés, celui de Roger Karoutchi mais aussi tout ce qui touchait aux ressources. Publicitaires qu'est ce que nous dit cet amendement,

Catherine Morin-Desailly. La, la suppression de la redevance, telle qu'elle a été faite l'année dernière en tout cas avec des solutions de remplacement qui n'étaient pas. Suffisamment travaillé et fait que aujourd'hui on revient un peu un point de départ et il faut réfléchir de nouveau sur la question du financement de de l'audiovisuel. Qu'est ce que nous dit également cet amendement c'est que. Ceux qui croient ce qu'il pensent ce qui XP espère. Que la pérennisation du système de de fraction de TVA par une modification de la LOLF et est un vote acquis, manifestement il ne l'est pas, puisque un certain nombre de. De signataires de cet amendement issu de la majorité sénatoriale montre que. La la le système de fraction de la TVA ne fait pas l'unanimité et qui la budgétisation est un scénario envisageable. Personnellement je ne partage pas. Je suis même en en désaccord mais ce débat telle que la présenter fort bien le rapporteur dans quelques instants. Il ne faut pas le minimiser. Et je me tourne vers vous Madame la Ministre parce que j'imagine aussi que ce débat entre pour schématiser entre budgétaire et. Ceux qui tiennent à ce qui est une ressource fiscale autonome. De nature fiscale autonome de de l'audiovisuel public, vous les retrouvez aussi au gouvernement entre Bercy et vous. Et on voit bien que tout est lié finalement le débat sur les ressources publicitaires et celui sur la budgétisation, on voit bien que le lien, il est très étroit, c'est-à-dire que on peut très bien imaginer que ceux qui tiennent à un système de budgétisation tiendront aussi à ce que l'audiovisuel public augmente ses recettes propres et en en particulier ses ses recettes. Publicitaires donc s'ouvrent maintenant un chantier qui va être complexe qui va nécessiter aussi un accord ici au Sénat, comme un accord à l'Assemblée nationale et je ne peut que rappeler à Madame la Ministre que cet accord ne pourra se trouvait que signer une vision partagée non seulement sur les ressources mais aussi sur l'organisation et la gouvernance. Merci. Il y a monsieur qui demande la parole est ensuite Madame, la ministre de. Je vois qu'on négocie. Sa. Le prochain mode de financement de l'acceptation de la Holding bon c'est du marchand de tapis tout ça. En réalité là, sur cette question de la redevance. Je suis d'accord vraiment. Presque en tous points avec ce qu'a expliqué Catherine Morin-Desailly. je ne suis pas d'accord avec vous Madame la Ministre sur la façon dont vous. Sous-estimez. Le fait que le mode de financement. Est directement liée à la question de l'indépendance de l'audiovisuel public.

Qui n'est plus parmi nous. J'aurais aimé que vous écoutiez son plaidoyer là-dessus. À la création de la redevance. Ça a été conçu et vécu comme un actionnariat populaire. Comme une participation directe ce lien Direct. Était très important. Et pourquoi Bercy s'acharne. Depuis. Que je suis sénateur et que je suis ses affaires. À vouloir. Empêcher ce lien Direct. Parce que Bercy n'aime pas. Que des ressources publiques lui échappe. C'est-à-dire que qu'il soit obligé. Là où c'est décidé. Il veut pouvoir disposer chaque année de. Ce pouvoir de négociation. Alors qui peut être pour des raisons d'équilibre budgétaire et cetera, c'est pas forcément la pression politique mais c'est insupportable. Et c'est ça qui a assuré l'indépendance. Et tous les personnels de l'audiovisuel public ça tous les acteurs de la création qui. Se sont mobilisés sur cette question, vous avez sous-estimé vous avez proposé un système avec la TVA qui va être caduque. Vous le savez au 1er janvier 2025. Monsieur Karoutchi propose une solution. Mais c'est ça on vous avez averti. Vous ouvrez la voie la budgétisation c'est la pire des solutions, parce que là c'est chaque année que ces renégocier et c'est Bercy qui donne le la. Et donc c'est pas la solution. Il faudra revenir sur cette question de la redevance. Merci de. Regardez ce qui se passe en Europe. Merci monsieur Assouline. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, justement, regardons ce qui se passe en Europe, 1 à Morin-, Desailly monsieur Assouline. Tous les pays n'ont pas une taxe affectée est-ce que l'audiovisuel public espagnol danois. Belge n'est pas indépendant, il est indépendant ça je je veux dire le mode de financement. C'est évidemment important pour garantir de la visibilité de la pérennité. Mais ça ne suffit pas à garantir l'indépendance, on le sait bien, on le sait très bien, sinon, quid, effectivement des pays qui ont budgétiser. Et d'ailleurs je je m'en réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 12 août 2022 qui a validé le dispositif de financement alternatif à la redevance en l'assortissant d'une réserve d'interprétation ayant pour effet de mettre à la charge de législature, l'obligation de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l'établissement de disette public soient à même d'exercer les missions de service public qui leur sont confiées. Donc le Conseil constitutionnel a posé une exigence relative au niveau de financement non à ces modalités. Voilà donc c'est, c'est assez clair et je pense que quand nous aurons de nouveau ce débat. Nous aurons en tête aussi tous ces éléments. Je vous remercie. Bien merci nous allons passer au vote sur cet amendement pardon, excusez-moi madame, Il est retiré. Bien il est retiré. Donc nous n'allons pas passer au vote et nous allons passer. Aux deux amendements suivants qui font l'objet d'une discussion commune. Madame Robert, non elle Suleiman. Alors monsieur Assouline le 39 oui. Alors c'est un amendement ou j'en parle souvent de celui-là. Qui va à l'inverse de ce qui est. Proposée par les uns ou par les autres. Chacun est attentif au fait que le service public puisse continuer à diffuser du sport puisse garder les manifestations qui l'a aujourd'hui qui permette de rassembler le peuple oui autour de grands événements. Il y a le Tour de France il y a Roland Garros. Qu'est ce qui reste d'autres. Le tournoi des Six-Nations. Déjà Roland Garros erronée. Je le répète. Il y a une hypocrisie totale à dire aujourd'hui que France Télévisions si elle en avait les moyens. Est libre d'acheter des manifestations cher le football et cetera y compris aujourd'hui. La Coupe du monde féminin qui n'a pas preneur. On verra s'il y a une suite. Et pourtant c'est un prix beaucoup plus bas que les prix. Ligue des champions et tout ça mais c'est déjà trop. Personne ici ne soutiendrait que ce soit de l'argent public et dans les caisses de ce qu'il faut monter les droits de façon incroyable, donc France Télévision est évincé. Parce que la seule façon de pouvoir acquérir ces droits, c'est d'avoir de la publicité au moment de ces manifestations. Pas un média. Ne peut se permettre d'acheter. S'il n'a pas la publicité pour payer. Donc le service public est puisqu'il a plus de publicité après 20h. Par contre, s'il avait les moyens d'acheter, c'est là que je pointe l'hypocrisie. Guy. Il y aurait de la publicité sur les maillots tout autour du stade sans arrêt qu'il ne reviendrait pas. France Télévisions qui reviendrait aux organisateurs. Mais ça serait autorisé. Ça serait autorisée. Par contre est interdit qu'à la mi-temps, il y a un spot publicitaire. Qui reviennent à France Télévisions. Donc c'est pas la publicité, le sujet c'est d'empêcher, France Télévisions et le service public d'avoir cette possibilité donc je repropose quelque chose que je proposais dans mon rapport. Sur le sport à la télévision que m'avait commandé le gouvernement. Je propose. Qu'après 20h, il puisse y avoir des spots publicitaires. En cas de manifestations sportives en Direct. Si bien sûr en Direct. Ensuite en discussion commune l'amendement 78 monsieur Fischler. Oui, monsieur le président. C'est dans la suite de ce qu'a dit. Notre collègue Assouline. C'est de rompre reprendre aussi un petit peu cette hyprocrisie qui fait que. Le sport pourrait passer entre 20h et 6h avec. Des des des marques publicitaire sur les maillots sur l'environnement du stade et qu'il ne puisse pas y avoir de publicité. Pour pouvoir justement on a dit. Souligne payer ses, ses retransmissions. Et moi je pense qu'il devrait y avoir une dérogation. Pour autoriser la publicité entre 20h et 6h, uniquement sur les événements qui sont des affichages déjà de publicité qu'on ne peut pas empêcher c'est simplement être moins hypocrite et permettent d'ailleurs donner les moyens à l'audiovisuel public de présenter ce type d'événement. Monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. S'agissant de l'amendement 39 de notre collègue David Assouline France Télévision dispose des moyens importants pour conserver des droits de diffusion sportifs sur ces chaînes le budget alloué par exemple à sa grille de programmes et le double de celui dont dispose TF1. Le groupe public a insisté pour obtenir l'exclusivité de la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. Pour plus de 130 millions d'euros alors que les chaînes privées étaient volontaires pour partager les coûts et les diffusions le rétablissement de la publicité en soirée dans les émissions sportives permettrait à France Télévisions de récupérer une quinzaine de millions d'euros par an. Cette somme peut être comparé aux 80 millions d'euros gaspillés en pure perte dans Salto, France Télévisions a davantage besoin d'une stratégie cohérente que de crédits supplémentaires. S'agissant de l'amendement 78 de notre collègue Bernard filles à l'air. Cet amendement vise à rendre possible la publicité en soirée sur les chaînes de France Télévisions lors des retransmissions sportives. Le groupe public a évalué à une quinzaine de millions d'euros les recettes que pourraient que pourraient rapporter cette disposition à comparer avec le montant de ses recettes publicitaires actuel qui atteint 380 millions d'euros et le montant de sa dotation publique qui s'élève, je le rappelle, à 2 milliards 8 d'euros. Cette disposition et donc anecdotique et ne permettra pas de financer l'acquisition de droits sportifs importants elle envoie par contre un signal négatif concernant la dépendance accrue du service public à la publicité et le risque d'affaiblir sa spécificité sur les deux amendements. Monsieur le Président, avis défavorable. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Cette fois, je suis totalement en accord avec. Que vient de dire le rapporteur. Je suis vraiment, je pense qu'on a un un point d'équilibre aujourd'hui qui est le qui a le bon la modération de la présence de la publicité sur les chaînes du service public. Ça fait partie Ça fait partie de cet élément de différenciation pour. Qu'il est important pour les Français qu'il convient de préserver. Et je pense que c'est pas le moment de déstabiliser les équilibres du marché publicitaire et. On, on connaît aussi les contractions de ce marché pour les chaînes privées, je pense qu'on a le bon point d'équilibre aujourd'hui avis défavorable. Il y a donc un double avis défavorable sur ces deux amendements. Je vais les soumettre aux voix. Monsieur Assouline. Madame la ministre a. Qui jusqu'à présent ne n'argumente pas trop puisqu'elle est contre tout mais là la. Argumenté et donc je vais lui réponde parce que. Non c'est pas vrai. Dites-moi. Là il y a un cas concret. Il y a la Coupe du monde de football féminin. C'est pas rien. Et l'équipe de France. En plus, on dit qu'il faut promouvoir le sport féminin. L'offre qui est proposé fait que peut-être. J'espère pas. Ce ne sera pas diffusé. Parce que aucune chaîne en clair n'est candidate. Voilà un. Un endroit où France Télévisions. Pourrait se positionner parce que c'est l'intérêt général. Parce que dans ses missions. Spécifiques citoyenne d'intérêt public, il faut favoriser le sport féminin. Et que c'est une compétition tout à fait importante. une copie une possibilité de publicité, même si c'est sur des faibles volumes. France Télévisions aurait pu se porter acquéreur toute de suite. Et il y aurait pas de sujet. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça va pas être fait, je, j'ai entendu, je ne sais pas vous avez peut-être vous en savez peut-être plus parce que ça devient une affaire publique qu'il y aurait une espèce d'offres conjointes entre M6 et France Télévisions pour y aller, j'ai lu ça ce que c'est vrai, pas vrai. Savoir que l'équipe de France féminine est en préparation. Que cette compétition arrive et qu'il y a aucune retransmission. De prévu parce que ça coûte trop cher est un scandale. Et là, le service public aurait pu candidaté s'il avait les moyens. Après 20h de faire une fenêtre publicitaire. Voilà donc c'est une réponse concrète à une. À des propos un peu trop généraux que vous avez formulée Madame la Ministre. Donc nous allons passer au vote sur ces deux amendements. Qui est favorable à l'amendement. 39. Le 1er de ces deux amendements présentés par monsieur Assouline qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement de monsieur l'air qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté et l'amendement 76 rectifié monsieur Fiole air. Ah oui. Donc je défendais la publicité entre 20h et 6h. Pour les événements sportifs, où il y avait de la, de, Justement de la publicité indirecte sur les maillots des environnements des des stades mais en revanche. Par cet amendement. La présence importante de parrainages de messages d'intérêt général et de publicité générique entre 20h et 6h sur les antennes nationales d'outre-mer et les plateformes de France Télévisions conduit à une situation regrettable. Où le téléspectateur a l'impression que la règle d'interdiction de la publicité sur le service public télévisuel entre 20h et 6h et largement contournée et nuit à la spécificité du service public de l'audiovisuel. Donc ce présent amendement vise ainsi la suppression de toute présence des annonceurs entre 20h et 6h sur les antennes nationales d'outre-mer et les plateformes de France Télévisions sauf campagne bien sûr d'intérêt général. cette interdiction serait notamment étendu à la publicité numérique et au parrainage. Excessif afin de réaffirmer l'objectif d'une diminution progressive de la publicité. Sur Sur toutes ses formes sur les antennes télévisées du service public et de conforter la logique de service public échappant aux logiques commerciales et d'anti-ici et d'anticiper la migration progressive des principaux annonceurs vers les supports numériques. Cet amendement perdre permettrait ainsi à l'audiovisuel de renouer avec l'esprit de la loi du 5 mars 2009 et de commencer plus tôt les programmes de soirée avec une totale liberté éditoriale. Avis du rapporteur sur cet amendement. Cette proposition figurait dans le rapport adopté l'année dernière par la mission commune des commissions de la culture et des finances sur le financement de l'audiovisuel public. Nous y sommes donc favorables sur le principe. En revanche, chers collègues. Il nous semble préférable d'évoquer globalement les moyens de l'audiovisuel public qui doivent être définis en fonction de ses missions. L'interdiction du parrainage sans compensation, aurait pour conséquence de mettre en difficulté le groupe public. C'est pourquoi il nous a semblé préférable d'instaurer un plafonnement des recettes de publicité et de parrainage dans la convention stratégique pluriannuel qui pourra commencer par stabiliser le montant de ces recettes avant d'engager leur baisse, à mesure que ses recettes alternatives pourront que des recettes alternatives Madame la Ministre. La. Merci monsieur le président, avis défavorable également pour ne pas. Revoir les équilibres qui nous semble bon aujourd'hui s'il y a des contournements du parrainage c'est à l'Arcom de de le vérifier. À ce jour en tout cas nous c'est le statu quo qui qui nous convient. J'en profite. Juste pour revenir sur le sujet de la Coupe du monde de foot féminin. Juste monsieur Assouline pour vous rappeler que comme elles se passent en Australie avec le décalage horaire on verra les matchs le matin donc le sujet de la pub après 20h. On ne va pas tellement aidé dans ce cas précis pardon j'avais oublié de dire sa tutelle. Bien. Nous allons passer au vote sur cet amendement pardon monsieur Fiole. Juste rappeler que j'avais proposé la compensation donc de ces pertes de recettes dans mon précédent amendement mais vous en avez pas voulu donc voilà où on se retrouve dans quelle situation se retrouvent.

Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté après l'article 5, un amendement 97 madame de Marco. Merci. Cet amendement a pour objectif d'instituer un conseil des auditeurs enfin de renforcer les Liens avec des sociétés audiovisuelles publiques. Il vise à instiller un peu de démocratie participative dans leur gouvernance sur le modèle de ce qui existe déjà. Au sein de la BBC. Ce conseil des auditeurs aurait pour rôle de participer au contrôle de l'application des contrats d'objectifs et de moyens ou des conventions stratégique pluriannuel au cas où. Et de la bonne application des missions de service public. Le Conseil aurait ainsi le pouvoir de saisir l'Arcom en cas de manquement constaté. Pour sa composition. Il faudrait que celui-ci celle-ci tiennent compte de la représentativité des auditeurs dans l'audience des chaînes concernées. Merci monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Il existe déjà des groupes et des associations qui rassemble des auditeurs. Par ailleurs, la loi Bloche a créé au sein de chaque chaîne des comités indépendants qui peuvent être. Il n'apparaît donc pas utile de créer une nouvelle structure qui n'aura pas une valeur ajoutée évidente c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur totalement d'accord avec ses arguments. 2 avis défavorables je soumets l'amendement voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons aux amendements qui concernent l'article 6. Avec 2 amendements en discussion commune qui sont des amendements de suppression le premier monsieur Bargeton. Défendu. Et le second madame monsieur Amendements de suppression. Le. Défendu. Et le 3ème excusez-moi il y en a trois. Madame de Marco. Toujours dans cette logique d'opposition à la Holding, nous proposons la suppression de cet article coordination enfin qu'il ne reste plus rien. Rien ne justifie cette réforme de de Villiers le public. Je voudrais rappeler les très bonnes audiences enregistrées en 2022 par Radio France qui reste le 1er groupe Radio France. À 30,3% de part À 30,3% de part d'audience et France Inter, la première radio niveau inédit de 12,6% d'audience. France Télévision est également en bonne forme, avec une audience cumulée de 29,4%, France 2. TF1 suivie de France 3. Dans ces conditions satisfaisantes entreprendre une réforme de rapprochement risque de fragiliser cette dynamique qui s'est installée et qui pour l'instant réussi au service d'audit audiovisuel public. C'est pourquoi nous nous y opposons. Merci monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Ce sont des amendements de suppression c'est donc un avis défavorable. Défavorable, madame la Ministre. Merci monsieur le président. À l'inverse ce sont. 3. Avis favorable. Donc, avis défavorable de la commission favorable du gouvernement je les soumet aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 6 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Nous passons l'article 7. Avec des amendements de quatre amendements de suppression. Monsieur Bargeton Merci monsieur le président. Bon c'est transformation de de l'INA en société anonyme pour qu'elle puisse intégrer la Holding. Alors évidemment ça peut paraître rien ça peut paraître simple et cetera mais ça montre ce qu'on voit depuis le le début, notamment l'article 5, c'est toutes les conséquences pour créer une Holding notamment la. De transformer public en société anonyme, ça veut dire énormément de ceux qui travaillent. Ça veut dire des transformations. Conséquente, de même que ce qu'on a vu sur le budget c'est c'est ça ça traduit en en pratique la consommation de temps et d'énergie que nécessitera la constitution d'une Holding au moment où on se consacre à la reconduction des. Des, des contrats d'objectifs et de moyens. Merci monsieur Assouline. Et juste en préambule. Madame la Ministre, vous avez raison sur les heures de diffusion. J'avais pris ça en cas d'école. Je vais ne va pas vous parler. Quelque chose qui est plus palpable. C'est ce qui se passe avec Roland Garros et les matchs la nuit maintenant rapt est capté par Amazon qui seule peut diffuser la nuit et vous savez que ça va aller en s'accentuant parce que ces. La nuit rencontrent du succès. La couverture l'éclairage le nouveau public. Et la et donc cette, ce, ce bastion on va dire du service public en terme de sport et menacée, vous le savez très bien donc voilà c'était j'avais cherché une illustration mais dont acte pour votre marque pour cette Coupe du monde là j'espère quand même que France Télévisions ou en tous les cas une chaîne en clair je je préférerais que ce soit le service public. Diffusera la la Coupe du monde féminin. Maintenant c'est une question qui est devenue politique. Cet amendement que je défends rapidement. S'oppose aussi. Par coordination à la création de la la Holding avec l'intégration en son sein, de l'INA. Une logique incroyable. Quelle est la logique d'intégrer l'INA. La Holding. Ce n'est pas un diffuseur contrairement aux 3 autres concernés les un établissement en charge de l'archivage des émissions de la numérisation de leur commercialisation et de formation qui joue un grand rôle dans la formation avec des missions particulières quand même la mise sur pied de l'école de la 2ème chance Alpha. Quelles synergies vous voulez trouver en intégrant cette. Société cette épique avec la radio. Ou la production et la diffusion d'informations et de fiction constituent les principales activités, je ne comprends pas la la logique. De parler de synergies et donc d'intégrer l'INA. La Holding. Madame brûlant. Nous nous opposons aussi à la transformation de l'INA qui est aujourd'hui un Epic en société anonyme. Pas seulement parce que ça va mobiliser des tas de juriste pendant quelques années, mais surtout parce que les épis, qu'ils ont été imaginés. Précisément pour porter des activités publiques de nature commerciale ou industrielle comme l'indique le nom des Qui ne pourrait pas être assumés par une entreprise privée soumise à la concurrence. Et il nous semble que c'est précisément ce qui définit l'INA. Qui. N'est rien moins que l'entité qui est chargée de protéger d'archives et de valoriser.

Mais c'est permettre qu'à la moindre, la moindre difficulté financière. Un acteur privé rentre au capital avec peut-être. Des intérêts qui seront éloignés de l'intérêt historique patrimonial et qui est développé par l'INA. et et c'est. C'est les les les chantiers dans lequel ils s'engagent. Montre qu'on est loin de la caricature que on fait parfois de des des entreprises de l'audiovisuel public puisque une date média a par exemple été créés au service des chercheurs qui a une offre de streaming qui se développe et qui est de plus en plus apprécié et donc il nous semble que l'INA doit évidemment garder son caractère des pics. C'est une sorte de protection de l'activité tout à fait exceptionnel et. Particulière que mène cet institut merci. Madame de Marco. Merci monsieur le président. Difficile également de comprendre cette proposition de changement de régime juridique. De l'INA, certainement, à mon sens une tentative de rationalisation budgétaire. Depuis sa création en 1974 a rempli des fonctions particulières au sein de l'audiovisuel public conservation des archives recherche de création audiovisuelle et formation professionnelle. L'INA est en outre dépositaire de dépôt légal à la radio et à la télévision depuis 1992. Au début des années 2000. La numérisation des archives est devenu un outil pour le développement de sa nouvelle stratégie commerciale de valorisation de tenu. Cela lui a permis par exemple de contacter. Contracté un accord avec YouTube en 2022 1011 et de bénéficier de recettes publicitaires. Jusqu'à la création d'une plateforme de streaming spécifique Madeleine. L'article 7 de la proposition de loi vise à le faire évoluer le statut juridique en société anonyme. En fin de l'intérêt à la Holding dans le dans un plus grand ensemble est qu'il est à craindre que les programmes développés par l'institut se trouve fragilisée comme sa plateforme. Merci monsieur le rapporteur. Avis sur ces amendements. Bien sûr. Merci monsieur le le président avec ce ce sujet de la formation et de l'INA, là on touche à quelque chose qui est caricatural. D'abord, chers collègues. C'est une demande expresse de l'INA. Répéter en audition. Et aujourd'hui, ils sont obligés de se soumettre aux règles là pour le coup une usine à gaz. La demande expresse de l'INA, c'est d'intégrer au contraire cette Holding et ça permettra certainement enfin à ce qu'il y ait une vraie coordination parce que là quand on parle de coordination. Je vous garantis, on n'en est pas on est loin du taux plein d'avoir l'ensemble des formations du service public à. Avis défavorable sur les quatre amendements. Madame la Ministre. Merci monsieur le président étant défavorable à la Holding je serais favorable aux amendements de suppression mais ça me donne l'occasion de rendre hommage au travail formidable qui est menée par l'INA et qui sans réorganisation sans mécano institutionnel a déjà avancé dans énormément de coopération notamment avec France Télévisions Lumni. France Info aussi avec Radio France. Sur la formation avec notamment les classes Alpha où j'ai pu rencontrer les jeunes en formation et là il y a aussi des avancées considérables. Donc. Bien évidemment, pour poursuivre cette priorité accordée à l'INA et à son développement mais favorable à la suppression de l'article 7. y a donc un avis défavorable du rapporteur favorable du gouvernement je mets aux voix les les amendements qui est pour. Et contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Je ne vois l'article 7 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Madame la Ministre, mes chers collègues. Il est minuit. Je vous propose de poursuivre encore un petit peu au maximum jusqu'à minuit et demi pour avancer un peu. Dans l'examen de ce texte, s'il y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. Donc nous passons à l'article 8. Avec quatre amendements identiques. De suppression monsieur. L'article

Oui. Je vais essayer de décrire le processus pour montrer à quel point. Les choses. Ressembleront une usine à gaz. Si cette loi venait à, à se mettre. En place. Donc la Holding, sera effectivement créée le 1er janvier 2024. Alors que le financement provisoire de l'audiovisuel public par une pension TVA aura encore cours. Qu'on sera sur un mode de financement. Au 1er janvier 2024, création de la Holding. 1er février 2024. Désignation de, de représentants des salariés des 2 personnalités indépendantes. Mi-février 2024 approbation par décret aux mise en conformité des statuts des sociétés concernées. 1er mars 2024 au plus tard, désignation des membres du CA de France Médias issu du Parlement, et des administrateurs et personnalités relevant du gouvernement ainsi que du représentant de l'État. Jusqu'au 1er janvier 2025, les présidents des quatre actuelle société son DG transitoirement ce qui les empêche donc a priori de devenir président de la Holding. 1er janvier 2025, entrée en vigueur du dispositif d'information du Parlement sur la part de ressources publiques affecté à France Médias et sa répartition des sociétés pour elle-même. Je ne sais pas comment va fonctionner une structure qui débute sur le thème basse très franchement. L'usine à gaz. Je pense que le terme est même faible ce calendrier de déploiement plus que complexe nous conforte dans notre volonté d'éviter la création de la Holding.

également souligné le risque que ce texte fait peser sur les salariés de la filière de l'audiovisuel public. La situation des éditeurs et éditrices contribuant matinales filmées, France Bleu, France 3 en grève depuis une quinzaine de jours illustrent les conséquences concrètes pour les salariés que que conduit la recherche perpétuelle d'économie en effet pour lancer ces matinales filmées émettre les images des journaux et radios. Il a fallu recourir à des éditeurs visuel au lieu d'embaucher ses journalistes, Radio France et France Télévisions ont fait le choix de sous-traiter ce travail en le confiant à une entreprise de production privée Eden presse au nombre aujourd'hui de 31. Ils sont employés en CDD eu ils n'ont pas de prime de précarité, pas de congés payés, pas de prime de matinale sont sous-payés mais en plus Eden presse viennent de signifier à celles et ceux d'entre eux qui ont cumulé trois ans de travail, que leur contrat ne sera plus renouvelé à la rentrée prochaine sachant que l'une des motivations de la création de cette Holding et de faire des économies, il y a fort à craindre que celle-ci ne conduise à de nouvelles suppressions de postes. Plus largement, cette Holding ouvrirez à terme la possibilité d'une fusion. Et avec elle une harmonisation des différentes conventions collectives des salariés des différentes sociétés de l'audiovisuel public. De nombreuses personnes sont concernées. France Télévisions représentant un effectif moyen de 9000 personnes. Radio France l'INA. etc les bonnes conditions d'exercice du travail des journalistes sur le corollaire de leur indépendance et je crains que cette Holding Bien précarisés terme celle-ci. C'est pourquoi nous voterons contre cet article par cohérence avec nos propositions de suppression de la Holding. Merci madame de Marco. L'article 8 prévoit les conditions de mise en oeuvre de la création de la Holding France Médias. Par cohérence bien sûr, nous proposons de le supprimer. Pourquoi ces dernières années, on constate un renforcement de la guerre de l'information et l'intégration de stratégie médiatique dans les stratégies de nombreux États cherchant étendent leur zone d'influence. Je pense à la Russie à la Chine mais aussi à l'Arabie Saoudite. Là aussi nos chaînes publiques ne mérite pas, comme le montrent les performances numérique de France 24 dont la chaîne YouTube quand même atteint 13 millions d'abonnés et RFI, qui rassemble 2 millions de monnaie toutes chaînes confondues. Cela illustre également la recherche de coopération et de synergies déjà à l'oeuvre et qui doit se poursuivre avant qu'un nouveau changement de structure soit envisagé. Cela montre également que les acteurs publics ont su se saisir des outils numériques pour se réinventer et qu'une verticalité excessive pourri nuire. Merci Monsieur le Président, par cohérence, ce sont des amendements de suppression donc nous y sommes défavorables. Madame la Ministre. Monsieur le Président, par cohérence, avis favorable aux suppressions. J'en profite pour vous rappeler comment. France Télévision est devenue France Télévisions, rappelez-vous. Loi de création de la Holding France. Télévision en août 2000. Entreprises unique en 2009 9 ans pour arriver à l'entreprise unique fusion des rédactions, France 2, France 3 2018. 18 ans après la loi. Holding et. Je relisais le rapport de 2016 de la Cour des comptes qui. Déplorait l'absence de synergies et d'économies. Donc ça veut dire qu'en plus cette. Hypothèse que à terme, il y aurait des économies ne ne marche pas. Voilà juste à. Rappelons-nous ce qui a déjà eu lieu et je vois pas en quoi aujourd'hui ça irait plus vite et ce serait plus simple. merci donc amendements de suppression avec un avis défavorable de la commission favorable. Du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adopté un amendement soins présenté par monsieur Merci Monsieur le Président c'est un amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 3 concernant les modalités de désignation du président de France Médias par l'Arcom. Bien qu'il a vite Madame la Ministre. Avis défavorable en cohérence avec tout ce que j'ai dit précédemment, mais favorable à réaffirmer la situation actuelle et nomination par l'Arcom. Bien je soumets l'amendement, on voit qu'il est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il est adopté. Je soumets aux voix l'article 8. Donc il est pour l'article 8. Qui est contre. Il s'abstient il est adopté. Nous passons l'article 9 avec 4 amendements de suppression. Bargeton. Défendu. Je suis Assouline. Non, madame Robert. C'est simplement, Monsieur le Président. Un amendement de coordination qui supprime l'applicabilité des dispositions de la Holding et de la loi du 30 septembre modifié dans certains territoires et pays d'outre-mer.

monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président, avis défavorable pour ces amendements de suppression. Madame la Ministre. Avis favorable. Donc, avis défavorable de la commission favorable du gouvernement. Qui est pour cette ces amendements. Qui est contre. Qui s'abstient et ne sont pas adoptés chou mets aux voix l'article 9 qui est pour. Et contre qui s'abstient-il être adopté. Avant l'article 10 l'amendement 81. Rectifié. Madame accord. Merci Monsieur le Président. Alors cet amendement de ma collègue Toine. Vise à clarifier les conditions de mise à disposition et de distribution des services de télévision. Les fabricants de terminaux radioélectriques connecté directement à Internet en vue de fournir une offre de services de communication audiovisuelle et exerce dorénavant une activité de distributeur de services ils établissent des conditions des relations contractuelles avec des éditeurs et des distributeurs en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle et propose désormais un univers de prescription et une éditorialiste façon des contenus alors que leur activité initiale pouvait être assimilée à celle de magasins d'applications, l'offre aujourd'hui proposée par les Smart TV et donc identique à celle des autres distributeurs de services. Par conséquent, ils doivent être assujettis aux mêmes obligations cet amendement de clarification vise ainsi à s'assurer que ces acteurs sont bien reconnues comme des distributeurs de services au sens de la loi du 30 septembre 1986. Cette modification corrige une asymétrie réglementaire en alignant les obligations entre toutes les formes de de distribution télé dans l'intérêt du public et des créateurs français face aux évolutions du secteur audiovisuel. Merci monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Cet amendement vise à considérer les fabricants de téléviseurs connectés comme des distributeurs, ce qui est le cas puisqu'ils organisent l'accès au service des éditeurs de programmes et des plateformes indépendamment des box et du signal diffusé par la TNT cette qualification permettra de leur imposer des règles similaires à celles qui s'imposent déjà aux distributeurs de type FAI ou Canal Cette disposition est donc au coeur des objectifs poursuivis par la proposition de loi afin de réduire les asymétries qui pénalise les chaînes c'est un avis favorable. Madame la Ministre. Merci monsieur le président. Alors votre proposition d'amendement vise, il me semble, a qualifié les constructeurs de téléviseurs connectés de distributeurs de services de télévision. Mais c'est déjà possible. L'article 2 1 de la loi de 1986 permet déjà au CSA devenu l'Arcom de considérer comme distributeur de services. Les constructeurs de téléviseurs qui nous des relations contractuelles avec des éditeurs, en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle, l'asymétrie réglementaire que que vous pointez ne me semble pas exister votre amendement se présente comme une clarification mais au fond il pourrait introduire en doute car il ne rappelle pas que pour être distributeur il faut établir des relations contractuelles avec un éditeur. Demande de retrait pour ma part. Bien, donc un avis favorable de la commission, une demande de retrait. Il est retiré. Merci. Donc nous passons à l'article 2 amendements sur l'article 10, monsieur Assouline. L'amendement 41. Oui pour comprendre, il faut situer l'intérêt. Vous savez donc que j'ai, j'avais été missionné par le gouvernement en 2016 pour revoir la liste des événements majeurs ce qui doivent être diffusés en clair. Qui procède d'un décret le dernier datait de 2004, il était un peu caducs et il fallait le moderniser. Donc j'ai travaillé longuement pour arriver à une proposition. Première question, madame le ministre. Est-ce qu'on va voir le bout, je sais pas combien de a eu depuis. Et et de ministre des Sports et de ministre de la Culture plus ça relève des deux. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire où ça en est. La principale innovation, je vais en parler tout à l'heure dans ma proposition puisqu'on me disait qu'il avait déjà trop d'événements. Et j'envoyais pas beaucoup de féminin. Je me suis dit, mais comment. Je peux réduire si en plus je peux pas ajouter les événements féminin j'avais proposé que tous les événements puissants tentent de façon équilibrée à compétition équivalente masculine. Il y a. L'obligation pour les compétitions féminines, ce qui serait une avancée très très importante dans la promotion du sport féminin et sa reconnaissance. Est-ce que vous pouvez me dire où on est le décret. Est-ce que cette mesure principale que je proposais a été retenu. Et puis là dans cet amendement c'était. La volonté de faire entrer quelques sports individuels populaire qui. N'étaient pas mis à l'honneur que les sports collectifs dans cette liste et notamment le Vendée Globe par exemple la Coupe de l'America. Les championnats de judo n'était pas dans cette liste pourtant. Il y a. Une baisse des licenciés dans les sports individuels et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aussi considérer que les sports collectifs dans les disciplines. D'importance majeure. Voilà donc. C'est cet amendement et là tu ensuite. Ce sera sur la question de l'équilibre entre le sport masculin et féminin. Et monsieur Assouline. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, cette disposition avait déjà été adopté au Sénat c'est l'article 9 bis dans le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux Oeuvres culturelles à l'ère numérique. Le débat avait alors permis de clarifier la situation sur le plan juridique, la définition de la liste des aînés des événements d'importance majeure ne relève pas du domaine de la loi d'autant plus que cette liste doit être notifié à la Commission européenne opère un contrôle strict. On peut ajouter qu'il n'y a pas nécessairement de modèle économique qui permettrait de diffuser en clair le Vendée Globe ou la coupe de l'America, avis défavorable. Monsieur le président. Alors je suis complètement d'accord avec le rapporteur techniquement. Cette proposition d'amendement ne relève pas de la loi puisque c'est un décret mais sur le fond. Je suis totalement d'accord avec les propositions que vous aviez fait et réitérées depuis 2016 et je comprends votre lassitude, monsieur le sénateur, parce que c'est long. Mais nous y sommes presque. En fait là nous a, nous travaillons sur l'argument. Ailleurs pour chaque. Fiche d'événements. On va passer d'une liste aujourd'hui de 21 événements d'importance majeure à une quarantaine et déjà on avait la liste la plus longue d'Europe. On va notifier tout ça. La Commission européenne. Mais vous savez qu'il y a un groupe de contact des États qui se réunit qu'une fois par an ça sera en décembre donc rendez-vous en décembre. Non, normalement on devrait arriver au bout. À ce moment-là. En tout cas sur le fond bien sûr, on va, on a repris plus de sport féminin plus de sport, on est complètement d'accord sur le fond.

Oui, bien entendu je je vais le retirer, parce que je sais qu'un décret, c'est pas une loi. C'était une façon de permettre ce débat et de poser ces questions à Madame la Ministre donc je retire cet amendement. Mais je défendrai quand même le suivant. Peut-être je le retirerai aussi. Bien merci donc. Ensuite il est retiré. Donc nous avons 2 amendements en discussion commune ensuite le 1er Madame de Marco. Non mais écoutez, moi je compte pas le retirer dès la Commission nous avions pointé l'obsolescence du décret du 22 décembre 2004, établissant la liste des événements sportifs majeurs et nous avions proposé qu'il soit réécrit sur la base de critères plus actuel. On peut s'étonner par exemple la faible part de compétitions féminines qui figure. Mais également de l'absence de la mention handisport. Enfin, le maintien du Grand Prix de Formule 1. Parmi les 21 événement donc. Paraît en décalage avec les aspirations actuelles de la société. Pourquoi ne pas y faire figurer d'autres sports un moindre effet sur l'environnement. Il est donc proposé de réécrire l'article 20 tiré de de la loi de 1986 et 2, confiée conjointement à la rédaction du décret au ministre chargé du sport et de la lutte contre les discriminations. Et l'amendement suivant monsieur Assouline. Oui donc c'est c'est un amendement qui va dans, dans le sens de ce que j'ai plaidé auparavant dans mes propositions de 2016, donc il y avait cette idée de créer une équité entre les les manifestations sportives présentes dans le décret. D'un des événements d'importance majeure féminin et handisport C'est une vieille. Déjà, proposition qui j'espère fera son chemin ou déjà j'ai une indication puisque Madame la Ministre je me dis qu'on est passé à 40. Donc forcément je me dit c'était avant donc ça a doublé. Donc ça veut dire qu'on a fait rentrer le féminin, et on se rapproche de de ma proposition. Merci de cette indication. Mais c'est vraiment important, il faut comprendre l'enjeu. De cela, il faudra réfléchir et ça peut être. bien sûr c'est pas la loi c'est un décret mais vous voyez bien que on est devant un sujet avec la Coupe du monde de foot féminin auquel on n'a pas de réponse On dit ça doit être diffusée en clair. Donc c'est obligé, même si une chaîne payante achète elle doit le sous-traité à une chaîne en clair si c'est diffusé. Mais il y a pas d'obligation d'achat. Ça veut dire qu'un événement qui ne trouvent pas preneur ne sera pas diffusé. Et donc il faut peut-être imaginer quand même parce que ça veut dire que si un jour les matchs de l'équipe de France sont trop cher, hé bien ils. Ne seront pas diffusée parce que les chaînes payantes n'auront pas le droit de de les diffuser. S'il n'y a pas une chaîne en clair qui le diffuse, c'est ça le principe des événements majeurs. Et on se retrouvera dans une difficulté peut être. Ça va venir assez vite. Cette histoire parce que c'est de plus en plus cher et il peut y avoir à des par moments aucun preneur là par exemple la Coupe du monde. Je viens de me rends compte que si il y a pas de preneur, c'est parce que c'est à midi et que peut-être le public qui va regarder est évaluée trop peu timbres important par rapport au coût.

Merci monsieur le président. On ne peut dénier une certaine pugnace cité à notre collègue David Assouline sur le sujet, ça c'est clair. Mais le gouvernement vient de commencer la notification du nouveau décret relatif aux aux événements d'importance majeure à la Commission européenne et il n'apparaît donc pas opportun de modifier les modalités de rédaction de ce décret. Sauf à prendre le risque de retarder d'au moins un an la sortie du nouveau décret ça c'était pour le l'amendement 94 rectifié, monsieur le président. S'agissant de l'amendement. Numéro 42. Je vais me répéter un peu mais comme pour le précédent amendement, le débat a déjà eu lieu dans le cadre de l'adoption de l'article 9 terre à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux Oeuvres culturelles à l'ère numérique. Il apparaît peu opérationnel de fixer des critères qui ne pourront pas s'imposer à la Commission européenne lors de l'examen qu'elle opérera de la liste des événements d'importance majeure c'est un David défavorable sur les deux. Il y a un double avis défavorable. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, avis défavorable également mais mais oui monsieur Assouline. Je vous confirme qu'on a bien pris en compte plus de visibilité pour le sport féminin et pour les. Le para sport les disciplines paralympiques. C'est complètement dans le sens de vos propositions justes aussi. Pour information, la Commission européenne comment elle va évaluer Toussaint de de 4 critères sont respectés, il faut que l'événement est un écho particulier dans l'État membre qui participent à l'identité culturelle nationale que l'équipe nationale y participe. Si c'est un sport collectif Que cet événement fasse traditionnellement l'objet d'une retransmission sur une télévision gratuite mobilisant un large public ça les critères il faudrait qu'il en ait au moins deux soient respectés. Donc ça va être analysé. Ligne à ligne pour chacun des événements qui seront proposées. On n'est pas encore complètement au bout mais on on y est presque. merci donc un double avis défavorable sur les deux amendements. Oui monsieur Assouline. Pour la même raison que tout à l'heure j'ai provoqué le débat mais je sais que c'est un décret donc je vais pas le laisser dans un amendement dans une loi. Merci. On a pas mal de précision. J'en ai plus que depuis plusieurs semaines en quelques minutes donc c'est pas mal et d'ailleurs il y a beaucoup de journalistes qui ont lieu. Écouter attentivement parce que il m'interroge et je ne peux pas leur répondre à ces questions. Donc ils ont les réponses et et c'est bien, c'est plus transparent. Merci merci votre amendement et est retiré. Madame de Marco, vous maintenez le vôtre. Oui. Donc, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 40 monsieur Assouline.

Monsieur le Président, la question de l'accès à des extraits avaient déjà été soulevés lors du débat sur le projet de loi relatif à la régulation et la protection de l'accès aux Oeuvres culturelles à l'ère numérique. Le débat porte une fois de plus sur le fait de savoir quelle doit être l'équilibre entre l'information du public et la liberté commerciale, il ne semble pas que le fait d'accorder aux chaînes gratuites, la possibilité de diffuser des courts extraits et de nature à mettre en danger le modèle économique des ligues. Cette disposition permet en outre de préserver l'attractivité des chaînes de télévision. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable. Madame la Ministre. Monsieur le président. Cet amendement. Oblige les ligues professionnelles a réservé aux chaînes en clair le droit diffusée dans leur émission des extraits des compétitions et manifestations qu'elles organisent. Les services de télévision peuvent déjà diffusé des extraits des compétitions sportives dont les droits ont été acquis par d'autres, c'est l'article L. 337 7 du code du sport. Tel qu'il est rédigé cet amendement va en réalité plus loin parce qu'il impose aux ligues d'attribuer un lot dédié pour ces chaînes en clair dans le cadre de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Ça me semble constituer une atteinte un peu disproportionnée à la liberté contractuelle pour ces raisons je suis plutôt défavorable à cet amendement. Un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. L'amendement suivant le 43 monsieur Assouline. La loi du 37 tombe 86 dans son article 22 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillent au respect par les services de télévision des dispositions concernant les événements d'importance majeure. L'article 9 du décret du 22 décembre 2004 a quant à lui précisé que saisie par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rendre un avis sur les conditions d'application des dispositions du décret. En réalité, le rôle du CSA n'est pas. Très précis. Précisément déterminée dans la phrase dans la phase de négociation. Sa capacité à rendre un avis notamment en raison des délais courts de négociations entre les éditeurs du payant et du gratuit. Il lui est difficile d'intervenir en amont en tant que tiers de confiance conciliateur arbitre des négociations jusqu'à récemment à faire Mediapro, en particulier, la réglementation des événements majeurs c'était impliqué de manière assez peu conflictuel et le CSA n'avait pas eu à formaliser Davy otite du décret de 2004. Il semble néanmoins qu'il y ait au moins un exemple dans lequel on peut considérer que le CSA en jouant un rôle non officiel de médiateur a contribué à la fixation du prix d'une transaction particulièrement tendue. Si les conditions de négociation des achats et des recettes de droits concernant les événements majeurs, continuer à se durcir. Il serait sans doute nécessaire de clarifier, de façon formelle au rôle du CSA en cas de conflit dans les processus de rétrocession notamment à sa capacité d'arbitrage final en cas de nécessité de vérification de la réalité de la retransmission au clair de l'intégralité des événements majeurs et de la possibilité d'appliquer une sanction en cas de non respect de cette obligation. Notre amendement prévoit ainsi que l'Arcom pourra adresser une mise en demeure au service ne respectant pas cette obligation de diffusion en clair des événements majeurs et en cas de récidive leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus. Vous voyez peut-être ou ça vous paraît technique mais si une chaîne. Payante Payante à événement majeur, elle est obligée de le vendre. Et de le, de, de le sous-louer quelque part à une chaîne au Caire. C'est le principe de l'avènement majeur, il doit être en clair et gratuit.

Merci, monsieur le Président, l'article 10 prévoit déjà un dispositif efficace pour obliger les plateformes à respecter la réglementation sur les l'événement d'importance majeure puisqu'il ne leur sera pas

Madame la Ministre. Oui même avis que le rapporteur mais mais je comprends la passion avec laquelle vous vous défendez ces amendements sur les événements d'importance majeure parce qu'au fond il s'agit de continuer à permettre à ce que ces grands événements sportifs fédère le plus largement possible nos citoyens. Mais là en l'occurrence là. Com dispose déjà d'un pouvoir de sanction. Après une mise en demeure préalable qui peut aboutir à une amende et on a les mêmes doutes sur la compatibilité avec le droit européen donc demande de retrait. retrait. Demande de retrait monsieur Assouline. Vous voyez, pour vous dire que les 15 secondes de dépassement. Tout à l'heure. Je vous fais économiser les deux minutes d'explications de vote. Je ne retire pas mais je ne vais pas plus loin dans dans la réponse. Bien merci. Donc, je le soumets aux voix avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement suivant monsieur Assouline 44 rectifié. Et toujours cette défense du sport à la télévision. Une instance de concertation suivi entre les différents acteurs du sport et de l'audiovisuel permettra de mettre à plat l'ensemble des problèmes qui grève actuellement l'attribution des droits télé et de préparer les filières aux mutations à venir, cette instance de concertation réunirait les organisateurs de compétitions sportives fédérations et ligues les éditeurs de services de télévision et de radio et les représentants de l'ensemble de la filière sponsors annonceurs et autres intermédiaires éventuellement publics, telle la ANS l'agence de moyens du secteur du sport. Cette instance s'inspire de la sport récréation une alliance instance créée dès 2005 lors de l'obtention par la ville de Londres de l'organisation des JO de 2012, grâce à laquelle ou cas sport la British Olympic Association et le comité d'organisation des Jeux ont établi une concertation avec l'ensemble des médias audiovisuels, non seulement pour favoriser la meilleure couverture couverture des épreuves notamment par les chaînes publiques, mais aussi pour favoriser l'assise populaire de cette manifestation qui a connu un grand succès. Parmi les questions qui pourraient être abordée par la commission pour ainsi figurer, celle d'un partage équitable, y compris au profit des au profit des diffuseurs des nouvelles sources publicitaire qui pourrait se développer dans l'avenir comme la publicité virtuelle pendant les retransmissions dans les enceintes. Le périmètre de l'instance pourrait être élargi à d'autres questions tu as de l'Exposition médiatique des disciplines et des pratiques sport féminin. Boire à l'ensemble des questions touchant aux relations. Sport et médias je. Dis pourquoi cette proposition. Étaient présents dans mon rapport de 2016, c'est parce qu'après avoir auditionné 50 fédérations et ligues je me suis rendu compte que. Chacune des fondée bien légitimement ses intérêts mais qu'il y avait aucune instance ou pour parler de cela, de droits de retransmission, elles étaient toutes ensemble pour chercher à dégager l'intérêt général. Donc elles étaient tous dans des B2B pour négocier leurs propres intérêts qui devenait contradictoire avec les autres et c'est important qu'il y a une instance où l'ensemble cherche l'intérêt général. En se réunissant avec les diffuseurs. Merci. Avis du rapporteur. Merci Monsieur le Président, l'expression usine à gaz a souvent été employé ce soir.-là, nous sommes en l'espèce devant un spécimen. Il n'apparaît pas nécessaire de créer un organe permanent pour conduire une concertation sur la retransmission des compétitions sportives un tel organe n'existe d'ailleurs pas pour le cinéma ou les séries. Par ailleurs, rien ne permet d'assurer que les participants. Accepteraient de siéger et qu'ils arriveraient à un accord, c'est le rôle du gouvernement, voire du Parlement de conduire une telle concertation en lien avec le milieu sportif et l'Arcom. C'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Même avis que le rapporteur finalement pourquoi le sport et pas d'autres secteurs. C'est effectivement une lourdeur supplémentaire et l'comme d'ailleurs associe d'ores et déjà les fédérations sportives, les acteurs du sport. À chaque fois il mène les consultations requises. Le comité national olympique et sportif français et cetera, avis défavorable. Il y a un double avis défavorable monsieur Assouline. c'est. Moi, une usine à gaz que votre ligne. Monsieur le rapporteur. Parce que c'est une instance qui peut se réunir, même une fois par an mais qu'il y a un moment où tout soit là. Et comprennent que. Eh bien il y a l'intérêt de l'autre et que les les corporatismes de sport particulier et puis aussi que les éditeurs et face à eux des acteurs et qu'on puisse discuter par une espèce de conférence annuelle. Des consensus qui peuvent se dégager faire progresser des choses notamment par exemple l'Exposition du sport féminin ou du handisport ça aurait permis d'avoir aussi des instances. Dessus, donc moi j'ai ressenti ce besoin quand j'ai fait ces concertations. Et ça n'a rien d'une usine à gaz, c'est beaucoup plus simple que la Holding. Si donc un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour cet amendement. Qui est contre. S'abstient. Il n'est pas adopté et enfin dernier amendement monsieur Assouline. Même si je crois qu'on a un peu traité le sujet mais le 45. Cet Cet amendement, conclut la série des amendements concernant la liste des événements d'importance majeure et il constitue une position de repli. La liste de ces événements issus du décret du 22 décembre 2004 est obsolète. Ah ne permet pas une représentation satisfaisante de très nombreux événements qui devrait être considéré comme majeur eux aussi et à ce titre, diffusé en clair et gratuitement pour en permettre l'accès au plus grand nombre de nos concitoyens. Le sport féminin d'abord des-t-il pas invraisemblable que la Coupe du monde féminine de foot qui a débuté dans à peine plus d'un mois n'est toujours pas trouvé de diffuseur et dans d'autres États européens, pas seulement en France, un en Espagne, en Italie, dans des grands pays de football des-t-il pas anormal qu'hormis le championnat d'athlétisme handisport aucune obligation de rentrer de retransmission de sports paralympiques en clair n'existent n'est-il pas anormal que Ligue pro ne soient pas tenus de réserver à des chaînes gratuites, des lots constitués d'extraits significatifs de leur manifestation et de leur compétition n'est-il pas normal que les sports individuels, hormis le tennis et l'athlétisme et le cyclisme ne figure pas dans cette liste comment réglera-t-on la question des plateformes de streaming qui ne sont pas contraints pas à l'obligation de diffusion clair. On nous annonce depuis longtemps la révision de cette liste Madame la Ministre nous a donné des indications mais qui sont à peu près celle que j'ai de. Puis 7 ans ça va bientôt arriver ça lui et ont nié. Donc maintenant. Je serai probablement d'ailleurs plus sénateur quand ça arrivera. Parce que ça va arriver très vite pour moi mais je. Soumets cet amendement. Comme une façon. D'insister. Merci monsieur le rapporteur. ne pourrait être réalisée en l'espace de six mois compte tenu du temps indispensable pour mener les échanges avec les autorités sportives et les délais nécessaires à la notification du décret. Auprès des instances européennes, c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Oui hélas, avis défavorable, parce que je je je comprends hein votre impatience. Je suis moi-même pressé de voir aboutir ce nouveau décret. Mais à terme, si moi ça marche même pas et que les délais de la commission là même si je disais qui se réunissent, qu'une fois par an, ce fameux groupe de contact pour discuter de ce décret. Mais là normalement en décembre si le dossier est complet si le groupe se réunit bien à la date prévue. Nous y arriverons. Et je vous emmènerai avec moi à Bruxelles, monsieur le sénateur.

c'était la Commission européenne qui l'aurait clamé qu'il fallait aller très vite, avant la fin du quinquennat de François Hollande. Donc j'ai fait ce boulot en trois, quatre mois, j'ai le jour et nuit parce qu'il fallait aller vite avec l'aide d'un inspecteur du ministère de la culture, excellent au demeurant je pense que je pouvais pas avoir mieux vous pouvez lui transmettre. D'ailleurs mes salutations s'il est encore là et qui avait fait ce travail avec quoi. Et puis patatras chaque ministre qui est venu derrière après 2017, culture, sport m'a dit. Ah. Oui, oui, on vient de m'en parler. C'est-à-dire qu'on lui avait pas transmis le dossier et puis quand il a, on lui avait transmis oui oui ça lui et c'est dans quelques semaines, vous vous rendez compte, 2016, on est en 2023 et vous me dites-vous maintenant que c'est en décembre bon bah de toute façon on prend mais c'est quoi ce fonctionnement bureaucratique fou. Qui est à contretemps de toutes les évolutions d'aujourd'hui et quand on nous dit que un décret est obsolète. Qui n'a de 2004 qu'on me le dit en 2016 et qu'en 2023 alors qu'on a on a on a donné les choses. Dans le détail, c'est-à-dire le décret, je l'ai écrit en détail. Eh bien on me dit bon. Bah. Je, voilà c'est c'est le fonctionnement français. Il rend pas optimiste sur l'organisation des pouvoirs publics et des décisions. Le monde va un peu plus vite que ça et on risque d'être dépassé. Si on continue.

Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le mardi 13 juin à 14h 30 pour les explications de vote, des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 et sur le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, la séance est levée.